La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point le procès verbal est adopté sous les réserves d'usage. Madame la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d'honneur des trois questeurs de la Chambre des conseillers du royaume du Maroc Monsieur Mohamed Salem Ben massage.

recollait Christian Cambon, président du groupe d'amitié France-Maroc est présent à leurs côtés, ils ont rencontré hier nos collègues questeurs du Sénat, ainsi que le président Roger Karoutchi et les membres du groupe d'amitié, la visite de nos collègues questeurs et le jumelage en cours entre nos 2 assemblées sur le reflet du partenariat qui nous unit et de l'importance, et j'y insiste, des relations d'amitié entre la France et le Maroc, madame la Première ministre, mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter au trois questeurs de la Chambre des conseillers du Maroc la plus cordiale bienvenue au sénat de la République française. Notre

Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement d'autres séances et retransmis sur Public Sénat. Demain. Et sur notre site. mes chers collègues, je vous rappelle la nécessité d'observer au cours de nos échanges, les valeurs qui sont essentiels pour nous, le respect des uns et des autres, et bien sûr aussi celui du temps de parole. Je donne immédiatement la parole à notre collègue Jacques Fernique, pour le groupe écologiste solidarité et territoires avait la parole. Monsieur le Ministre, la semaine dernière, madame la Première ministre présenter l'ambition France nation verte et vous y a fichier l'enjeu des mobilités, mieux se déplacer parmi les 6 thématiques d'impact Direct sur la vie des Français aux horizons 2030 et 2050, mais, mais, dès à présent en 2022 pour 2023 votre gouvernement se donne-t-il les moyens de ses ambitions pour les mobilités vertes au moment où nos transports publics du quotidien sont plus que jamais nécessaire qu'il s'agisse du ferroviaire de nos régions ou des transports publics urbains et ruraux, au moment où ils apparaissent, bon pour le pouvoir d'achat, bon pour la décarbonation bon pour la vitalité économique de nos territoires, ne risquons-nous pas faute d'engagement à la hauteur de laisser se dégrader ses services de compromettre les chances d'un New Deal des transports publics, comment ces services publics essentiels pourrait-il se maintenir ces prochains mois, sans encadrement des coûts de l'énergie sans plafonnement des prix de l'électricité ferroviaire comment nos trains régionaux et no futur réseau Express métropolitain pourraient-ils prospérer si les péages ferroviaires déjà les plus élevés d'Europe continue d'augmenter, comment nos transports publics pourrait-il s'équilibrer si le versement mobilité les employeurs et remise en cause s'il n'est pas confortée comment réussir un choc d'offre des transports urbains et l'électrification des bus comment enfin avec les moyens limités de votre projet de loi de finances moderniser hein ferroviaire français qui pourraient décrocher en Europe, monsieur le Ministre, quelle réponse concrète maintenant pour dégager l'horizon des transports publics et ferroviaires. On vous répond : la parole. Et comme ministre délégué en charge des transports, Monsieur le Ministre Monsieur Clément Beaune. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous avez raison d'insister sur le caractère absolument central du ferroviaire et les transports publics, notre ambition écologique de neutralité carbone pour 2050 transformation profonde de notre économie, notre société, la première ministre est l'occasion de le dire dès l'arrivée du gouvernement nous portons à Christophe Béchu, le ferroviaire et la colonne vertébrale de cette mobilité propre, le projet de loi de finances dont le Sénat aura à connaître dans quelques jours le démontrent déjà mais je tiens à le signaler, vous avez parlé d'ambition limitée, je ne vous rejoins pas sur ce point mais je précise une chose que j'ai l'occasion de dire devant votre assemblée en commission, c'est que le PLF ne retrace pas l'ensemble de l'effort public et de l'effort d'État en faveur des mobilités vertes et du ferroviaire en particulier, au total, ce sont pour 2023 et c'est un chiffre qui n'a pas été atteint depuis plus de 15 ans, un total de 12 milliards d'euros qui sont mobilisés par l'État 4 milliards d'euros directement dans le PLF il nous avons tour les efforts de la Société du Grand Paris, le budget de de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et beaucoup d'autres encore, c'est 12 milliards d'euros, dont la moitié plus de la moitié exactement seront consacrés au ferroviaire, nous avons besoin de poursuivre cette ambition, vous avez souligné à quel point nous devions entretenir notre réseau ferroviaire, le transport du quotidien, c'est l'ambition que nous portons à Christophe Béchu, que s'agissant du réseau ferroviaire français, je le dis depuis que je suis arrivé, c'est la priorité absolue, nous avons un contrat de performance qui a rehaussé de manière inédite, les crédits annuels pendant 10 ans que nous consacrons réseau ferroviaire français et nous augmenterons cet effort dès le PLF 2023 et nous attendons le Sénat il contribue d'ailleurs le rapport du conseil d'orientation des infrastructures pour voir ensuite quelles seront nos priorités qui seront déclinées dans une programmation actualisé dans les prochains mois en même temps que nous mettrons en place des contrats de plan État Région qui feront aussi une part très significative aux transports publics et aux transports ferroviaire, faut-il regarder d'autres options, travailler sur l'offre à baisser les coûts de l'énergie, comme nous sommes en train de le faire pour éviter qu'il y ait des difficultés en 2023, oui, nous y travaillons, aller comme ça que nous éviterons des difficultés sur l'offre dans les prochains mois et je suis prêt à regarder avec le Sénat, comme tout le gouvernement, l'ensemble des leviers que nous pouvons activé sur la base du rapport du dans les prochains mois. Je vous entends, monsieur le ministre, il y a vraiment urgence, le président du Grand-Est parle d'être contraint peut-être de fermer des lignes, on envisage ici ou là des hausses de tarifs, donc Monsieur le Ministre, agissez vite et fort pour contrer ces repli face à la crise, merci. La parole est à notre collègue Pierre-Jean hier Jelen pour le groupe, les indépendants, République et Territoires, vous avez la parole. Madame la Ministre, les causes sont multiples : déjà la guerre déclenchée par Poutine et ses conséquences sur l'approvisionnement en gaz, ensuite le manque d'anticipation et d'entretien du parc nucléaire qui fait qu'à l'heure où nous parlons, près de la moitié des réacteurs ne fonctionne pas et, enfin, un système de fixation du prix européen complètement dépassés, résultat des courses : le prix de l'électricité n'est plus maîtrisée, les ménages sont pour le moment plus ou moins protégé par le bouclier tarifaire, les commerçants, les usines, les entreprises totalement exposé il y a 2 jours, je voyais encore un boulanger qui avait payé l'an dernier 2500 euros de facture électrique, on lui propose pour l'année prochaine en 2023 des contrats qui approche 20000 euros juste intenable, les collectivités, pas de visibilité budgétaire qui va peser évidemment sur les investissements et sur les capacités à assurer les services du quotidien, il existe des dispositifs de soutien trop restrictif et trop complexe, il y a la réponse de fond quel mix énergétique pour quelle indépendance mais là maintenant, tout de suite, dans les jours qui viennent, nous avons besoin d'une réponse coordonnée à l'échelle européenne, et on peut dire que ça ne démarre pas très bien, un plan d'aide de 200 milliards mis en place par l'Allemagne qui est de nature à créer une concurrence déloyale, un sommet européen la semaine dernière qu'il n'a pas apporté les réponses attendues et un conseil des ministres franco-allemand qui s'est transformé en un déjeuner à l'Élysée, le temps presse, les entreprises, les collectivités doivent renouveler leur contrat avant le 31 décembre et elle s'interroge sur le thème je dois-je signer ou pas signer la proposition mon fournisseur d'énergie, madame la Ministre, pouvez nous nous dire où en sont les négociations avec nos partenaires européens et les mesures envisagées, merci. On vous réponde, la parole est à la ministre de la transition. énergétique Madame Pannier-Runacher vous avez la parole. Merci Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Vert Eulen vous soulignez à juste titre l'action du gouvernement pour protéger les ménages mais également les petites entreprises de moins de 10 salariés et les petites collectivités locales parce que je veux rappeler ici que le dispositif de bouclier énergétique que nous avons mis en place, il couvre les petites entreprises et les petites collectivités locales et il permet à ses petites entreprises à ses petites collectivités locales de bénéficier du prix de l'électricité, le plus bas d'Europe, alors vous avez raison, il faut aller plus loin, il faut aller maintenant travailler pour nos nos grandes entreprises et faire en sorte de trouver un dispositif et les autres collectivités locales qui ne sont pas couvertes mais vous savez que des premières propositions ont été faites avec un filet de sécurité pour amortir le choc de cette augmentation du prix de l'électricité pour ce faire, nous agissons au niveau européen, vous avez mentionné, monsieur le sénateur, le Conseil européen ce Conseil européen, il a t'arriver à un consensus de 27 pays sur des mesures très claires de coordination sur le prix du pour demander à la Commission de faire des propositions sur ce prix du gaz qui permettent d'installer un corridor et de contenir le prix du gaz sur le prix de l'électricité avec un découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité sur une plateforme d'achat commune du gaz et sur des mesures techniques, je dirais, mais très importante pour permettre de faire des coupes circuits sur le marché et marché financier d'échange d'électricité et de gaz, c'est une avancée majeure et c'est le président de la République, qui les a obtenus d'autre part, au plan national et vous le savez, nous travaillons avec Bruno Lemaire avec Christophe Béchu à mettre en place également une garantie, électricité et des aides qui soient appropriés à chacune des situations, vous savez que pour les PME, nous avons, a priori, un dispositif qui devraient les protéger partiellement et nous finalisons ces travaux, vous savez que pour les ETI et les grandes entreprises, Bruno Lemaire négocie actuellement une augmentation des aides du cadre, Ukraine et un relâchement des conditions pour en bénéficier, donc, tout ça me travaille avec 10 milliards d'euros dans le cadre de notre trajectoire budgétaire pour faciliter et la vie de ces entreprises.

Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, le gouvernement a finalement changé de politique et décidé de rapatrier collectivement toutes les femmes et les enfants de djihadistes retenus en Syrie pourquoi. Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, Mesdames messieurs. Les sénateurs, monsieur le Président, Chaouchi, je serais tenté par un parce que mais. je comprends parfaitement qu'il ne vous conviendrait pas, en réalité, nous n'avons rien changé nous rapatriant d'abord chaque fois que c'est possible en terme de sécurité pour nos agents qui, bien sûr, je veux rendre hommage, deuxièmement. Notre doctrine n'a pas bougé d'un millimètre, il faut que les femmes demandent le rapatriement, troisièmement, c'est une judiciarisation systématique et je tiens à vous indiquer que toutes les femmes ont fait l'objet d'un mandat de dépôt, sauf une, pour des raisons médicales, et puis il y a le problème des enfants. Au fond, s'agissant des femmes de la judiciarisation, elles ont choisi

il y a un devoir d'humanité et de vigilance humanité parce que ce sont des enfants qui n'ont rien demandé que ce sont des enfants français que comme le disent certains pédopsychiatres, ce sont des bombes à retardement qu'il faut veiller sur eux mais qu'il faut que nous le fassions parce que les laisser là-bas, c'est prendre le risque qu'un jour ils reviennent ici pour commettre des abominations et puis de voir évidemment de vigilance dans un suivi qui est pluridisciplinaire psychologiques, psychiatriques éducatif, je ne pense pas que nous ayons bougé d'un millimètre et d'ailleurs il y a quelques jours de cela, je me suis complètement exprimée devant la commission des lois du Sénat et Monsieur le Président, buffet a dit de mon intervention Jean Rosie encore qu'elle était claire et et si vous souhaitez davantage de renseignements, je vous suggère, Monsieur le Président, Karoutchi d'aller dire mon intervention. Monsieur le Président, Karoutchi. Monsieur le Ministre, les femmes qui demandent à revenir, elles le font parce que nous ne les avons pas déchu de la nationalité française, ce que le Royaume Uni, ce que le Royaume-Uni a fait à l'égard des djihadistes, ce qui lui permet de ne pas récupérer les gens retenus en Syrie, je me permets de vous rappeler également que lorsque Nicole Belloubet était garde des Sceaux en 2019, 2020, elle nous disait ici, hein, la France préfère qu'il y ait des jugements en Irak avec des tribunaux mixtes et ensuite, elle nous a dit, puisque ça n'est pas faisable dans tous les cas, nous ferons du cas par cas et nous ne ferons revenir en France

de rapatrier ses ses épouses de jihadistes et le président Macron à l'époque avait répondu : pas question, c'est beaucoup trop dangereux pour la sécurité des Français en quoi la sécurité des Français en 2022 est différente de celle de 2019 surtout, monsieur le garde des Sceaux et vous le savez, et c'est bien que la justice s'occupe des femmes qui reviennent, mais la plupart d'entre elles, la plupart d'entre elles ont continué dans les camps de détention en Syrie, sur les réseaux sociaux a vanter les mérites de Daech a vanté les mairies des attentats et du fait de pouvoir continuer la lutte des djihadistes en France et ailleurs, voilà qui nous avons fait rentrer. La parole est à notre collègue. Amel gars car, pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues, pour commencer, permettez-moi de saluer la mémoire des gendarmes, récemment décédé d'adresser une pensée aux familles et à leurs collègues ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition énergétique le groupe Imerys ça a annoncé la mise en exploitation minière d'ici 2027 d'un gisement de lithium dans l'Allier, qui sera l'un des plus grands d'Europe, ce qui est une bonne chose en effet le lithium connaît un essor considérable car indispensable à la révolution numérique et à la transition écologique, il est notamment nécessaire aux batteries des véhicules électriques, on estime aujourd'hui une augmentation des besoins au lithium de 42 pour 100 d'ici 2040 et certains experts craignent une pénurie d'ici 2030, il s'agit d'une bonne nouvelle, stratégique, d'abord pour notre souveraineté énergétique puisque nous dépendons aujourd'hui entièrement de la Chine pour nous approvisionner en lithium, l'annonce du groupe Imerys permet d'affirmer, à nouveau, que notre pays, l'Union européenne ont enfin besoin de mener une politique minière ambitieuse et responsable, le projet Emilie est également une bonne nouvelle écologique car il n'y aura pas de décarbonation sans électrification enfin autre intérêt du projet économique cette fois-ci, puisqu'il mérite évoque la création de 1000 emplois Directs et indirects dans la région, il ne s'agit pas d'un projet neutre je souhaite attirer votre attention et vous questionner sur la gestion des risques sociétaux et environnementaux qui accompagne cette exploitation, la consommation d'énergie, les rejets toxiques, notamment, sont fréquemment pointée du doigt d'après Imerys cette mine sera exemplaire sur le plan écologique et respectera le standard international Irma pour pallier à ses incidences bien sûr encore une fois, c'est une bonne chose, l'acceptabilité sociale de ce genre de projet n'est pas à sous-estimer, là où sont annoncés, les projets d'extraction minière des collectifs se constitue aussi, il y a nécessité à rassurer l'opinion publique en instaurant des normes respectueuses de notre environnement, mes questions sont les suivantes : comment le gouvernement compte-t-il accompagner le respect de ses engagements et l'acceptabilité l'acceptabilité pardon local du projet, la mine durable va-t-elle enfin voir le jour en France, merci. madame la ministre de la transition énergétique Madame Pannier-Runacher. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Guéquières merci d'abord de souligner combien ce projet participe d'une politique de transition énergétique qui anticipe, qui cherche à ne pas remplacer une dépendance aux énergies fossiles par une dépendance à d'autres matières premières critiques comme le lithium, le nickel et le cobalt et vous le savez, ce projet mairie s'il s'inscrit dans le plan France 2030 et il fait partie des 5 projets que nous soutenons pour justement recréer une chaîne de valeurs autour de c'est à métaux critiques qui seront absolument nécessaires pour la production de batteries électriques, et vous savez combien ça compte notamment sur notre territoire commun du Pas-de-Calais et plus largement des Hauts-de-France puisque nous accueillons la vallée européenne de la batterie électrique et nous aurons besoin de ces matières premières alors pour aller plus loin dans le cadre européen et dans le cas national, cela fait maintenant plus de 18 mois que nous travaillons à créer une filière responsable autour de ces métaux critiques autour de 3 actions sécuriser des approvisionnements à l'étranger, qui soient des approvisionnements dans des mines, et qui appliquent ce référentiel domine responsable qui est notamment portée au niveau de la Commission européenne par le vice-président Sefcovic deuxièmement, mettre en place toutes les actions de recyclage et ça fait partie des projets que nous soutenons, au niveau de France 2030 pour faire en sorte que toutes les matières qui rentrent sur le territoire français, d'une manière ou d'une autre puisse être réutilisé et justement ne pas avoir à devoir rechercher dans nos sous-sols des matières premières critiques et 3ème élément, en responsabilité, regarder la faisabilité de développement de de mines mais sur un registre domine Responsable partagée au niveau européen, il y a des cas de mines responsable je pense à celle du tungstène, en Autriche, qui avait été d'ailleurs présenté lors du conseil compétitivité à Lens que j'avais organisé autour de cette notion qui est au milieu d'un parc naturel et l'autre que l'on peut agir dans ce sens nous agirons donc dans ce sens en responsabilité au niveau européen et au niveau national. Merci l'apparence est à notre collègue Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, nous vivons une crise majeure de notre système de santé qui est à bout de souffle des urgences au service pédiatrique en passant par la neurologie, la psychiatrie, tous les voyants sont au rouge à l'hôpital public, sur l'ensemble du territoire personnel épuisé soignants qui partent, petit à petit, dégoûté par leurs conditions de travail dégradées depuis de longs mois 4000 professionnels en pédiatrie, viennent de lancer un appel au président de la République, dénonçant les conditions désastreuses de prise en charge des enfants transferts multiples affectations dans des services adultes non appropriée sortie trop précoce des programmations d'opération mise en danger de petits patients ce n'est pas la faute de la bronchiolite, mais bien de la politique : une menée depuis des années dans les hôpitaux, à coups de restrictions budgétaires successives et irresponsable des cris d'alarme se lancer régulièrement par des professionnels, notre groupe les relais ici dans l'hémicycle, vous les ignorez comme tous vos prédécesseurs face à l'urgence de la situation et la mobilisation des professionnels, vous avez dû annoncer le déblocage de 150 millions le un plan blanc et des assises de la pédiatrie au printemps, cela n'a convaincu personne dans la crise est grave et structurelle allez-vous enfin, autant d'appels de ces professionnels qui parle de perte de sens dans leur métier, conséquence de la gouvernance bureaucratique et de la tarification à l'activité allez-vous comme il vous le demande, rouvrir des lits dans les services de pédiatrie en arrêtant la fuite des soignants et en recrutant des jeunes qui sont passionnés. On vous réponde, la parole est au ministre de la Santé et de la prévention Monsieur Brown, vous avez la parole. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Cohen j'imagine bien sûr que je suis très près le problème de notre hôpital public, je le suis. Depuis plusieurs semaines en étant en contact d'ailleurs avec les professionnels de la pédiatrie que j'ai rencontré à plusieurs reprises, je le suis depuis que je suis arrivée au ministère et pour être honnête, je suis même depuis de nombreuses années pour suivre ces difficultés, vous avez annoncé un certain nombre de choses que l'hôpital n'allait pas bien depuis plusieurs mois, permettez-moi de vous dire que l'hôpital ne va pas bien depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, grâce, grâce ou à cause de politique comptable, je vous rejoins, dont un certain nombre ont été votés par l'ensemble du Parlement depuis malheureusement trop longtemps en ce qui concerne l'engagement de ce gouvernement en ce qui concerne l'engagement depuis 2000 17 du président de la République, ce sont 53 milliards d'euros qui ont été mis en plus dans l'hôpital pour répondre, certes à des problèmes conjoncturels mais également à des problèmes structurels à vous parlez de de la pédiatrie, des problèmes de de bronchiolite de quoi par le temps, nous parlons effectivement d'une épidémie de bronchiolite qui survient plus tôt qu'avant sur un hôpital qui est, vous l'avez dit vous-même à bout de souffle mais j'irai là aussi dans le dans le même sens, je tiens à saluer d'ailleurs au passage, mes anciens collègues et les soignants dans tous les services qui travaillent dans des conditions difficiles en ce qui concerne la bronchiolite qui est une pathologie qui est inquiétante, qui fait peur et je comprends l'inquiétude des parents, je veux aussi rappeler qu'elle est très majoritairement bénigne et doit être pris en charge en priorité par les médecins généralistes, alors les réponses qu'apporte son gouvernement sous l'impulsion de la première ministre des réponses structurelles avec un budget de 150 millions d'euros supplémentaires qui est mis pour répondre au problème aigu d'un certain nombre de services, ses services de pédiatrie bien entendu en en 1er recouraient, j'en profite pour rappeler que ce ne sont pas uniquement les urgences pédiatriques mais plus au niveau des services de pédiatrie et puis une réponse plus structurelle sur l'entame du système hospitalier en ce qui concerne la pédiatrie nous débutons dès la semaine prochaine des travaux pour aboutir au printemps et je l'ai annoncé à des assises de la pédiatrie qui nous permettront de prendre des vraies décisions structurelles sur ce secteur.

et que vos solutions ne sont pas bonnes, nous n'avons pas voté les Budgets austéritaire nous au niveau de notre groupe et qui mettent à genoux l'hôpital quand allez-vous rehausser réellement l'Ondam à la hauteur de l'inflation, vous ne le faites même pas pour 2023 vous n'écoutez pas les professionnels vous n'écoutez pas les parlementaires et vous dites tout va bien, ça va très mal et il faut vous agissiez en urgence qu'est-ce qu'il y a de pire que de trier des patients de choisir entre 2 enfants la responsabilité, elle est pas du côté des professionnels de santé, elle est du côté du gouvernement, et vous pouvez aussi la paix, nous rencontrons les professionnels, ils sont très en colère contre vous agissez. La parole est à notre collègue Julien Bargeton. Pour l'Europe, un groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Monsieur le président merci, ma question s'adresse à Madame la ministre de la culture, Madame la Ministre, la baisse du de fréquentation des salles de cinéma d'environ moins 25 % par rapport à 2019 inquiète les professionnels du secteur, d'autres évolutions comme la consommation des films ou des séries sur les plateformes à domicile les inquiète également si le cinéma français doit certainement se réinventer, il s'agit d'un système que nous devons préserver Simone Les harkis novembre un beau matin l'innocent, la rentrée montre la vitalité et la diversité et la singularité du cinéma français, son système repose sur la mutualisation, les films à succès finançant les films plus fragiles, n'oublions pas que le cinéma d'auteur est né en France dans les années 50 en réaction au cinéma américain plus industriel qui faisait appel aux têtes d'affiche, n'oublions pas non plus que les films dits du milieu qui font aussi la spécificité du cinéma en France souffre beaucoup. La photographie c'est la vérité et le cinéma, c'est la vérité, 24 fois par seconde, disait Jean Luc Gaulard, mais pour que cette vérité émerge, il faut le choix d'une mise en scène, il faut un chef opérateur ou une chef opérateur, il faut des comédiens, des comédiens, des dialogues écrits ou des silences, des ellipses, il faut de la qualité, Madame la Ministre, quelle appréciation portez-vous sur les évolutions en cours structurel ou bien conjoncturel quelles perspectives, pouvez-vous donner aux professionnels pour redonner l'envie aux Français de rejoint les salles obscures et pour garantir le financement de notre système unique merci beaucoup. Pour vous répondre, la parole est à madame la ministre de la culture Madame Abdul-Malak. Monsieur le président, Monsieur le Sénateur, Julien Bargeton, mesdames et messieurs les sénateurs. Merci de nous donner l'occasion de parler du cinéma en ce jour où nous lançons une campagne de communication pour soutenir les salles. On a tous une bonne raison d'aller au cinéma, je suis sûre que tous, ici, sur ces bancs, vous aurez votre bonne raison d'aller au cinéma, c'est une campagne pour mobiliser nos citoyens pendant un mois, c'est une campagne pour recréer du désir d'aller en salle, voir les films en grand au-delà de cette campagne de court terme, à plus long terme, je suis persuadé que nous avons tous de bonnes raisons de croire en l'avenir du cinéma. Pourquoi, parce que d'abord, la France reste une nation de cinéphiles, certes, nous avons perdu un quart de public par rapport à l'avant-Covid mais c'est bien pire ailleurs moins 60 % de fréquentation en Italie moins cinquante pour cent, en Corée du Sud, moins 40 pour % en Espagne ou en Allemagne, donc notre filière résiste et les Français restent cinéphile. Par ailleurs, l'État accompagne un élan nouveau, celui de la jeunesse avec le Pass culture 2 millions et demi de places de cinéma sont partie financé par l'État pour inciter les jeunes à aller au cinéma, 76 % des jeunes interrogés disent allaient plus au cinéma grâce au Pass culture la filière aussi grâce à elle, elle se réinvente, vous l'avez dit-elle restent très mobilisés dans les années 80 90 on nous prédisait la mort du cinéma à cause de l'avènement de la télévision, la fréquentation avait chuté à 110 millions de spectateurs et ça a doublé dans les années qui suivent et parce que la filière s'est réinventer parce que l'État était aussi à leurs côtés et je le précise, le soutien de l'État n'a jamais été aussi fort, il y a un arsenal de soutien pour soutenir cette filière du cinéma qui est unique au monde, déployés pendant la crise sanitaire 500 millions le budget du CNC pour le cinéma 100 millions de crédits d'impôts pour le cinéma et le plan France 2030, qui nous permet de déployer 350 millions d'euros aussi pour la filière je le dis à la jeunesse, il y a énormément de bons films à voir pendant les vacances de la Toussaint, vous qui êtes en tribune en famille venait, aller au cinéma, beaucoup d'émotion, vous attendent. Madame Madame la présidente, Laurence Rossignol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci monsieur le président, 11000. 11000 c'est le nombre de TER supprimés dans les Hauts-de-France depuis le 1er janvier 2022. 129 c'est le nombre de trains supprimés retirer dans les Hauts-de-France pendant les vacances de la Toussaint, au prétexte que les élèves n'est, en ne prenant pas le train, on peut retirer 129 trains demie, c'est le temps qu'on passait à la gare du Nord, la semaine dernière des usagers jusqu'à onze heures et demie du soir pour s'entasser ensuite dans le dernier train je vous parle des Hauts-de-France, je vous parle des trains supprimés vous savez supprimé c'est la malédiction qui tombe sur les voyageurs, quand ils arrivent dans les gares, que ce soit à la gare du Nord à Beauvais, à Lens, à Saint-Quentin, partout, je vous parle d'de France parce que c'est ma région, je pourrais vous parler tout aussi bien de toutes les régions de France, y compris l'Île-de-France monsieur le Ministre des usagers quotidiens du train sont des salariés, des gens qui prennent le métro, le train, le RER pour se rendent de leur lieu de travail, à leur domicile et ses salariés, ils prennent le train, parce qu'ils ne peuvent pas se loger là où il travaille, ou alors ils ne peuvent pas travailler là où ils vivent, ils ont accepté des emplois ou des logements loin l'un de l'autre parce qu'il y avait des transports collectifs, c'est essentiel dans leur mode de vie, c'est ce qui structure et qui détermine leur organisation de vie et l'imprévisibilité de transports publics désorganise totalement leur vie cette imprévisibilité elle mais leur emploi en danger, elle insécurisé parents qui ne savent jamais à quelle heure ils pourront aller chercher leurs enfants à l'école et j'ai une pensée toute particulière pour ces femmes qui, le matin, prennent le train à Creil ou le soir pour faire les, les, les ménages dans les bureaux, les conséquences sont multiples, maltraitances des voyageurs report sur la voiture, émissions de CO2 désorganisation du travail et de l'économie française, monsieur le ministre, il y a urgence, que faites-vous.

je partage d'abord les mots que vous avez eu pour les galères que vivent un certain nombre de concitoyens dans la région des Hauts-de-France mais aussi dans d'autres régions face à des difficultés spécifiques dans les transports publics, la priorité que j'ai décrite il y a encore quelques minutes, en réponse au sénateur Fernie qu'elle n'est pas théorique, nous avons augmenté les moyens cette année pour le réseau et pour les transports du quotidien maintenant pour répondre à une situation difficile, il faut nommer les choses de manière précise et que chacun assume ses responsabilités, de quoi parle-t-on de transport qui sont régionaux et donc il y a une situation spécifique aux de France que je discuterai à nouveau avec le président Bertrand j'ai évoqué d'ailleurs le sujet avec le prix n'aura pas ici même au Sénat il y a une semaine et il faut que chacun soit prêt à mettre les moyens nécessaires, la région en particulier qui a la responsabilité d'organiser les trains Express régionaux, il faut le dire, l'État sera là en soutien pour un certain nombre de projets, nous le ferons pour le réseau Express métropolitain, j'ai changé, par exemple avec le président Castelain, de la métropole pour que nous résolvions le problème : la livraison du train Alstom dans les prochains mois, donc nous agissons ce sur quoi nous sommes responsables et je veux le dire aussi, du côté de la SNCF, j'aurai une réunion avec le PDG de la SNCF en fin de semaine, parce que les questions d'offres qui relève sans doute de l'opérateur et je veux que l'État joue son rôle à plein qu'est-ce qui se passe, en particulier dans la région des Hauts-de-France car chaque situation est spécifique ou devons y répondent précisément il y a des pénuries de recrutements et donc il y a des difficultés, les suppressions pour les vacances que vous avez évoquées sont beaucoup lié à ça et donc je ne me résous pas à ce que nous vivions dans cette situation de cette manière pour les mois qui viennent, il faut accélérer les recrutements, la SNCF a lancé un plan exceptionnel de 440 recrutement pour la seule région Les Hauts de France pour les TER et donc en travaillant ensemble avec la région, avec ce qui relève de l'État avec l'opérateur SNCF nous améliorerons la situation, les prochains mois, vous avez raison de dire que c'est difficile, mais il faut que chacun puisse assumer ses responsabilités financières, d'organisation et de moyens. Merci, je vais donner maintenant la la parole notre collègue Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, vous avez la parole, mes chers collègues. Merci. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur Marc Fesneau Ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, monsieur le Ministre, les Français se sont découverts depuis quelques années un engouement croissant pour le tourisme en montagne un environnement au mode de vie si particulier, s'agissant de l'autre versant, celui de la vie montagnarde, la loi montagne a permis d'instaurer des politiques adaptées à la vie en altitude en matière d'agriculture, la loi pose ainsi un double principe celui général de la préservation de l'activité contre les contre les préjudices causés par les actes de prédation et celui de la régulation pour maintenir l'existence de l'élevage, si des mesures ont été mises en place, notamment après la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées en 2018 et la propagation du loup sur l'ensemble du territoire, le malaise des éleveurs persiste, tandis que les prédations continue, l'été dernier le loup était à peine identifiés dans le massif du Hautacam dans les Hautes-Pyrénées, quand relevé déjà 26 attaque pour 43 brevis tué, malgré la grande réactivité des services de l'État, que je salue et qui très tôt se sont tenus au côté des éleveurs, il en est de même dans l'Hérault en Lozère, dans les Alpes de Haute-Provence et d'un temps d'autres départements touchés de plein fouet par la prédation du loup aujourd'hui le problème des prédations perdure malgré les demandes de fortement relayée du Sénat face à l'ampleur du phénomène, l'association nationale des élus de la montagne, a adopté jeudi dernier une motion rappelant l'obligation de défense de l'agro-pastoralisme et une meilleure gestion des grands prédateurs, nous ne l'oublions pas l'agropastoralisme est une activité agricole d'excellence qui joue un rôle de régulation de la végétation et contribue au développement de l'activité économique et touristique aussi, Monsieur le ministre ma question sera simple quelles mesures nouvelles comptez-vous mettre en place afin de répondre à la demande des éleveurs dans l'activité pastorale continuent d'être menacés, nos éleveurs sont aujourd'hui à bout, ils attendent des dispose des dispositions et des décisions fermes et efficaces, je vous remercier. Or vous répond : la parole est au ministre de l'Agriculture et de la souveraineté. Alimentaire monsieur Marc fait de vous avez la parole. Merci, merci, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Carrère, je voudrais vous remercier de cette caisse de me poser cette question qu'pose la question de l'équilibre entre agro-pastoralisme et en particulier j'étais comme vous le savez, en fin de semaine dans le Doubs, puis dans sa voix, enfin dans les de sa voix pour évoquer en particulier cette question qui est très prégnante, nul ne peut évoquer cette question et vous avez raison de rappeler sans souligner quand on est auprès des éleveurs, j'ai été rencontré un éleveur qui venait d'être prédatés le sentiment de détresse, le sentiment d'impuissance et le sentiment d'incompréhension qu'ils ont de la prédation et de la menace que ça fait peser sur deux sur eux 2ème élément rappeler quand même que le pastoralisme, vous l'avez dit, pour des questions touristique, mais c'est un modèle qui est un modèle exemplaire aussi en terme de biodiversité, il y a besoin de préserver la biodiversité du lot, mais il a aussi besoin de préserver les autres formes de biodiversité qui sont garantis par les activités de pastoralisme et d'agriculture extensive, alors comment nous ne pouvons agir d'abord le président de la République l'a rappelé dans votre département, cet été, l'idée c'est qu'au niveau européen, nous travaillons sur le statut de l'espace, l'espèce à partir de données scientifiques 2ème élément, c'est que nous travaillons au niveau national, le président d'ailleurs à cette occasion, avait rappelé le développement d'une 2ème, brigade de loup pour travailler sur ces questions de prédation 2ème élément travail au niveau national sur quoi on peut travailler avec mon collègue Christophe Béchu avec Bérangère Couillard, nous travaillons sur ce sujet dans le cadre du plan national ou ou à l'extérieur de travailler sur des modalités de simplification simplification pour effectuer les prélèvements réellement simplification dans les procédures d'indemnisation trop souvent l'indemnisation ne tient pas compte de l'ensemble du préjudice qui est porté, on est que sur les animaux prédatés mais pas ceux qui sont perdus ou la perte génétique et ça c'est un élément qui est important 3ème élément travailler sur un dénombrement qui fasse l'objet d'un consensus, puisque c'est à partir de ce dénombrement que les prélèvements sont effectués 19 % de la population recensée enfin dernier élément, il faut qu'on travaille aussi sur le statut du Patou qui pose des tas de questions juridiques pour les éleveurs, évidemment, quand ils viennent mordre ici ou là, un touriste voilà madame la sénatrice, on est bien sur un chemin que nous entendons tracées avec mon collègue Béchu ma collègue Couillard pour avancer concrètement et donner des moyens pour avancer pour qu'on préserve l'agro-pastoralisme, on le doit aux éleveurs, ils vont le dos à la biodiversité, mais à toute la biodiversité, merci, merci, merci. Le ministre, la parole est à notre collègue Jean-Raymond Hugonet pour le groupe Les Républicains. Merci, merci, monsieur le président, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la culture depuis le 2 septembre dernier le groupe Canal Plus a cessé de diffuser les 5 chaînes du groupe TF1, à la suite d'un différend commercial concernant le renouvellement du contrat de leur distribution, la justice a eu l'occasion de se prononcer, à 2 reprises sur ce différend qui pénalisent tout particulièrement les foyers situés en zone rurale et en zone de montagne et qui reçoivent la télévision numérique par satellite, en considérant que la loi ne crée aucune obligation à la charge de Canal Plus de reprise des chaînes de la TNT et qu'aucun contrat écrit signé avec le groupe TF1 n'obligeait Canal Plus à mettre à disposition ses chaînes, la cour d'appel de Paris a certes clarifier la situation du point de vue du droit, mais elle n'a pas résolu les difficultés rencontrées par des millions de Français, le gouvernement est resté très discret depuis 2 mois sur cette situation, tandis que l'Arcom qui a proposé plusieurs fois sa médiation estime qu'elle n'a pas les moyens juridiques d'imposer un compromis dans ces conditions, que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour permettre aux Français qui ont sont aujourd'hui privés d'accéder à la TNT. Monsieur le président, Monsieur le Sénateur Hugonnet je partage vos préoccupations. Vous l'avez dit, cette situation résulte d'un différend commercial d'une négociation commerciale qui n'aboutit pas. Il ne m'appartient pas de m'immiscer dans cette négociation commerciale, mais en tant que ministre de la culture, je suis évidemment très attentive à l'accès de tous à l'offre gratuite de la TNT, j'ai dès le début de ce conflit, écrit au président du groupe Canal Plus pour en appeler à son sens des responsabilités de l'intérêt général pour éviter de priver des foyers des 2 millions de Français, de l'accès au aux 5 chaînes du groupe TF1, pour l'instant cette négociation n'a pas encore abouti, et effectivement, vous avez rappelé les décisions de justice, vous avez rappelé les déclarations de l'art comme une modification de la loi sera probablement à l'avenir, nécessaires pour éviter que cela se reproduise et que des téléspectateurs soit pris en otage de ce type de négociations nous y travaillerons ensemble, je l'espère en tout cas à court terme, je sais que les discussions ont repris, nouveau patron, qui est arrivé aussi à la tête de TF1 Rodolphe belle-mère avec Canal Plus, espérons collectivement qu'ils parviendront à un accord qui permettra de rétablir au plus vite l'accès aux chaînes gratuites de la TNT. Monsieur Gonnet. Madame la Ministre de l'adage dit que l'espoir fait vivre en l'occurrence, vous nous appelez à l'espoir, il ne s'agit pas d'espoir, la réalité est simple : la loi de 1986 qui a été modifiée, chers collègues, plus de 80 fois depuis 86 et qui sous-tend l'écosystème de l'audiovisuel est aujourd'hui à genoux, cette loi, votre collègue Franck Esther que je vois ici au banc également avait commencé à porter une réforme très rapidement, elle a été abandonnée aujourd'hui, elle a été abandonnée en rase campagne, pour des raisons de Covid qui était simple : à l'époque à mettre en avant la raison est ici au Sénat, nous sommes prêts à travailler sur cette loi de 86 revisité par ce qu'il faut se mettre aujourd'hui à jour des plateformes numériques et des usages des chaînes de télévision notamment, nous vous appelons à ce chantier, chère madame. La parole est à notre collègue Jean-Marc Todeschini pour le groupe socialiste, écologiste et républicain tout seul président les chers collègues, Madame la Ministre. Pendant que les médias français était occupé par le feuilleton du 49 3 à l'Assemblée nationale tomber les conclusions du sommet européen qui était à la limite de la débâcle pour la France et qui consacrer l'échec de 50 politiques européennes, françaises, projet phare du président de la République, les Allemands, une partie des pays européens ont fait prévaloir leur point de vue quant au prix du Taz et nous renvoie, nous les Français, à nos problèmes de maintenance de nos centrales nucléaires, l'accord de principe sur un bouclier antimissile entre plusieurs pays aux Européens autour de l'Allemagne sans la France se dans l'OTAN s'est félicité nous laisse, je dirais, isolé sur le concept d'une Europe de la défense, malgré le conflit en Ukraine sur le spatial, l'Allemagne s'oppose au principe de préférence européenne et développe seul en mer du Nord, des projets de Pascal dédié au micro lanceur force est ce constater le recul de notre influence en Europe et en même temps, la France se voit reprocher une certaine arrogance les dissensions dans le couple franco-allemand sont tellement importants qu'il a fallu pour la 3ème fois reporté le sommet franco- allemand qui devait se tenir aujourd'hui à Fontainebleau, ces multiples alertes doivent être entendus, l'Allemagne depuis le Brexit est au centre du jeu européen et regarde désormais plus à l'est et vers les Balkans que vers Paris, elle défend ses intérêts, elle s'affirme comme leader de l'Union européenne ou les pays du nord lui sont acquis depuis longtemps alors Madame la Ministre quelles leçons tire la France cette situation pour nous éviter un isolement sur le plan international et en particulier au sein de l'Union européenne. Pour vous répondre. La parole est à madame la secrétaire d'État chargé de l'Europe. Madame Laurence Boone, Madame la Ministre, vous avez la parole. monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Todeschini écoutez, nous n'avons absolument pas la même vision des choses, je vais commencer par vous. Les que nous avons tous des enjeux communs due à la guerre en Ukraine, qui porte sur l'énergie, qui porte sur la défense et qui vont ensuite porter évidemment sur d'autres domaines économiques, y compris le spatial. Ces enjeux communs, ils se reflète aussi avec le changement géostratégique, vous avez vu la position de la Chine et comment elle évolue tous les pays font face à ces gens, je mets pas de la même façon, quand c'était la crise du Covid c'était les économies de services qui étaient les plus affectées aujourd'hui quand c'est l'énergie, ce sont les économies manufacturière et l'Allemagne fait face à des conditions très difficiles d'énergie de fournitures, puisqu'il faut qu'elle en trouve ailleurs qu'en Russie, mais également de prix. Face à ces enjeux, qu'est ce que nous faisons, le président de la République pendant le Conseil européen a invité le président Charles crédit et à discuter ensuite c'est lui monsieur qui a réussi à unifier les positions pour que nous ayons un compte à un communiqué à la fin du Conseil, qui étudie absolument toutes les mesures énergétiques qui peuvent être spécifiques à chaque pays enfin aujourd'hui, ces problèmes cette défense, l'énergie et de réorganisation du monde, ils vont pas se résout dans un claquement de mains et c'est pourquoi le président a invité le chancelier Scholz à venir déjeuner et d'ici aux 60 ans du traité de l'Élysée, nous allons travailler ensemble pour pouvoir converger sur tous ces sujets, mais voyez-vous, ce sont des efforts qui demande plus que des paroles, des actions et du travail, je vous remercie. savais ce que Madame la Ministre, difficile pour vous de répondre, je dirais que tout va très bien madame la marquise, mais je vous rappellerai le discours du président de la République

au niveau de la réflexion français sur l'Union européenne, le président de la République avait utilisé pour l'OTAN, le terme d'encéphalogramme plat, j'ai peur qu'aujourd'hui on soit nous soyons nous réduit à un ça on les remplace dans le développement de l'Europe. La parole est à notre collègue Max Brisson pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, depuis, Aristide Briand la religion ne peut faire obstacle à la loi et la République a peu à peu, donner à la laïcité, une dimension singulière dans l'enceinte de nos écoles, pourtant le mois dernier, tout comme on publié les chiffres du chômage, vous annoncez monsieur le Ministre, Éducation nationale, 313 atteinte à la laïcité, mais Monsieur le Ministre, 313 atteinte à laïcité, ce sont en réalité 313 violation de la loi, à défaut de nous rassurez-vous s'affirmer n'avoir pas la main qui tremble, vous appelez que les équipes vous rappeler que les équipes valeurs de la République ont été renforcés, tout comme la formation des professeurs en fait vous annoncer un plan de communication sur les réseaux sociaux pour réduire l'action des influenceurs ne pensez-vous pas plutôt face à un projet politique radical, celui de l'islamisme qu'il faille et d'abord appliquer la loi dans toute sa rigueur, la semaine dernière, proviseur parisien disait Ahzoune interview collégiens qui fume, on le sanctionne des élèves qui portent des tenues religieuses, c'est plus compliqué, on manque de cadres précis alors Monsieur le ministre ma question est simple quand allez-vous donner à tous les chefs d'établissements de France, un cadre précis des instructions précises que pour que, face à ces violations de la loi, ils aient la certitude d'avoir le soutien de leur hiérarchie pour appliquer la loi, toute la loi, règle la loi. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Brisson en la matière, vous avez raison, la boussole, c'est la loi de 2004 et j'ai bien indiqué qu'il fallait une application ferme stricte de la loi de 2004, vous avez rappelé le renforcement des équipes valeurs de la République, nous parlons ici de plusieurs centaines de personnes à l'échelle du territoire nous les renforçons encore la formation, vous l'avez rappelé des sanctions ont été prises contre des élèves récalcitrants, elles seront encore prises au terme des procédures engagées, nous allons d'ailleurs vérifiez également relancer et préciser les choses en matière de sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion définitive des élèves concernés et, en effet, des sanctions de cette nature ont été prises, vous avez également mentionné la question des réseaux sociaux, c'est une question juridiquement délicate d'un point de vue pour s'attaquer directement à ses comptes et à ces influenceurs néfastes qui ne veulent ni de bien aux élèves ni de bien à l'école ni de bien à la République, mais nous sommes très actif là-dessus et je vais recevoir un certain nombre de dirigeants de ces réseaux sociaux pour les mettre devant les responsabilités, nous sommes et nous serons très actif et très vigilant sur cette question, enfin, la laïcité, c'est une question aussi de sanctions, j'en ai parlé vous avez mentionné en effet ce que j'ai dit je n'ai pas et je n'aurai pas la main qui tremble là-dessus, mais c'est aussi une question de pédagogie, nous avons une bataille à mener et à mener de nouveaux pour faire bien comprendre que la laïcité est une liberté la possibilité de transmission de savoir qu'il se fasse sans interférence, la garantie de l'émancipation et de l'éducation des futurs citoyens de la République. Monsieur le Ministre, je crains que vous ne répondiez pas au chef d'établissement, ils se sentent seuls, ils ne veulent pas avoir arbitré, ils veulent des consignes claires pour ne pas avoir à interpréter, ne les laissez pas seul votre collègue, Gérald Darmanin, parle d'une offensive islamiste visant les plus jeunes, elle passe par l'école, alors Monsieur le Ministre, préciser le cadre donné des instructions au chef d'établissement, soutenez-vous, chef d'établissement pour que désormais il soit assuré que toute violation de la loi soient sanctionnés. La parole est maintenant notre collègue Catherine Morin-Desailly pour le groupe de l'Union centriste. ma question concerne plusieurs ministères mais s'adresse à Madame la ministre de la culture qui a tutelle sur les collections publiques en juillet 2020 pour célébrer le 58ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, la France a restitué à Alger, 24 Khan, détenu au musée de l'homme, supposés être ceux de chefs de la Résistance tués pendant la conquête coloniale, or, une enquête du New York Times vient de révéler que la majorité des crânes ne serait pas ceux de résistants mais non identifiés ou d'origine incertaine, certains parlent d'imbroglio de procédure parfaite, d'autres de scandale d'État, il semble que le travail du comité d'experts scientifiques franco-algériens qui oeuvraient depuis 2018 à l'identification des crânes, condamné à la plus stricte confidentialité été écourtée, pourquoi, comment ce geste hautement symbolique de réconciliation que de côté sont nullement sur le fond mais sur la forme, le gouvernement ayant décidé du seul d'une convention de dépôt et non d'un acte législatif de restitution, tout en en revendiquant l'appellation pourquoi cela a été Madame la Ministre, le Parlement garants des collections nationales totalement coûtant des dans cette affaire et je le regrette, est en droit d'obtenir des réponses. Pour vous répondre, la parole est à madame la ministre de la culture Monsieur le président, madame la sénatrice Morin-Desailly, merci de votre engagement sur ce sujet, je sais que. Vous portez cet engagement de longue date et c'est un enjeu qui me tient très à coeur cette politique de restitution, c'est regarder notre histoire en face c'est nouer des relations de partenariat et d'amitié nouvelle avec d'autres pays, avec d'autres peuples c'est un chemin subtil respectueux qui a un chemin qui n'est ni celui du déni, ni celui de la repentance qui est celui de la reconnaissance, je voulais vous apporter quelques précisions sur le cas des crânes algériens qui ont été déposés et non pas restitué en effet les autorités françaises et algériennes ont mis en place en décembre 2017. Un comité mixte qui était chargé d'identifier formellement ses restes humains dans les réserves du il y a eu un travail d'étude rigoureux qui a duré 18 mois, la commission est arrivé à la conclusion que 24 crâne sur 45 remplissait toutes les conditions. Pour être restituées, mais c'est sur cette base consensuelle et documenter qu'ils ont été remis sous la forme d'un dépôt à l'Algérie, il n'a jamais été dit le contraire, d'ailleurs je vous renvoie aussi au communiqué final du du comité intergouvernemental de haut niveau qui précisait aussi ce terme de restes humains présumés algérien conservés dans les collections publiques françaises au paragraphe 19. Donc on avait pris toutes les précautions nécessaires sur ce sujet, au-delà de ce cas spécifique, et nous aurons l'occasion d'en reparler, nous allons travailler ensemble à des lois-cadres pour poser une doctrine, une méthode, des critères de restituer habilitées, pour qu'à l'avenir sur différentes catégories de sujet que ce soit les restes humains, que ce soit les biens spoliés juif un cas très différent ou que ce soit les biens pillés pendant la colonisation en Afrique ou pris de façon illégale ou illégitime, nous aurons de riche débat pour définir ces critères et une orientation qui pourrait être celle d'une loi cadre sur chacun de ces 3 sujets, je vous remercie. La Morin-Desailly. Je me réjouis, enfin de ce travail partagé le Sénat comme vous le savez, engager des travaux très importants avec mes collègues Pierre Ouzoulias et plusieurs autres collègues, le soutien de notre président de commission, Laurent Lafon, nous avons d'ores et déjà formulé des propositions et un texte de loi voté à la nuit, en janvier dernier, sur la question des restes humains dits sensibles, ce texte aurait été complètement votée, il aurait résolu complètement la question de restitution des crades à l'Algérie, au demeurant je vous madame la mise que malgré tout vous défendez l'indéfendable, car j'ai les conclusions là de la commission qui s'est réunie le 25 juin 2020, chargée d'examiner les propositions de restitution de ces restes humains d'origine algérienne et quelles sont quand même les conclusions de la commission, elle dit bien la commission alerte sur le risque de protestation sur le caractère précipité et autoritaire de l'opération, la Commission note que les modalités imposées par l'urgence diplomatique interrompre le travail de mémoire réalisé par le comité d'experts, et j'en passe, parce qu'il y a d'autres remarques qui souligne aussi que, et c'est fort dommage que le ministère de la culture culture écarté comme le Parlement l'a été, de cette procédure, je pense qu'il faut remettre de l'ordre dans ce sujet pour souligner l'importance du bien-fondé de la réconciliation des mémoires. Merci.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues se sont actuellement 6500 soignants en pédiatrie, qui ont signé une lettre ouverte au président de la République où il dénonce les mises en danger quotidiennes des patients dans des services saturés en cause l'épidémie de bronchiolite et des services hospitaliers très fragilisé qui peinent à recruter et à garder du personnel notamment paramédical, pourtant, l'épidémie de bronchiolite est habituel à l'Automne et donc prévisible, monsieur le Ministre, cette situation n'est malheureusement pas nouvelle en 2019 déjà, faute de place en réanimation des enfants ont dû être transférés hors de la région Île-de-France, mais aujourd'hui ce problème se pose avec acuité sur l'ensemble du territoire et des enfants sont régulièrement transférés d'un hôpital à l'autre, parfois même à plus de 200 kilomètres : comment en est-on arrivé là les capacités d'accueil des services se dégrade en raison de la fermeture de lits et de manque de personnel soignant, on manque de médecins libéraux ont restreint l'accès aux urgences et on ne fait plus appel au kinésithérapeute pour les bronchiolites, pourtant, d'après une étude, la plateforme a qui respire l'offre de soins en kiné respiratoire permet de réduire de 13 % les consultations pédiatriques au CHU de Bordeaux le week-end, toujours le même constat : le gouvernement n'a rien anticipé et gère la pénurie avait des rustines le déclenchement de plan blanc oblige à déprogrammer des interventions chirurgicales pour une simple épidémie de bronchiolite, sans qu'il y ait véritablement de perspective d'amélioration, vous avez annoncé le déblocage de 150 millions d'euros pour les services en tension à l'hôpital notamment pédiatrie mais Monsieur le Ministre est-ce que le gouvernement envisage enfin de mettre en oeuvre des mesures structurelles en revalorisant significativement la permanence des soins de nuit du week-ends et jours fériés en augmentant le nombre de pédiatres en libéral, et à l'hôpital et en acceptant que les kinés puissent à nouveau intervenir pour lutter contre l'épidémie de bronchiolite, comme c'était le cas auparavant. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé et de la prévention. le problème lié à la bronchiolite et à nos hôpitaux, vous savez que ça me préoccupe particulièrement, mais je veux apporter quelques précisions dans ce que je peux entendre non on ne trie pas les enfants à l'entrée de l'hôpital, les mots ont un sens, celui-ci s'est ajoutée artificiellement de l'inquiétude de l'angoisse aux parents, ça peut même être plus dangereux que ça, en poussant à du renoncement aux soins donc je je le redis avec force notre système de santé prend en charge tous les enfants en situation de détresse, système de santé dans son ensemble, il le prend en charge dans des parcours de soins identifié pour réponde aux besoins, je le redis, toutes les bronchiolites ne doivent pas aller à l'hôpital. Quel parcours vous parlez de la place des des kinésithérapeutes, il y a plusieurs mois, la Haute autorité de santé a relevé que certaines pratiques de kinésithérapie habituel faites sur la bronchiolite sont dangereuses qu'il faut les arrêter, donc la place est maintenant beaucoup moins importante, dès qu'il était un peu dans cette pathologie précise alors : où et comment savoir ou faire prendre en charge son enfant, lorsqu'on a une crise de bronchiolite à des difficultés respiratoires, hé bien, je le redis aux parents, si vous ne savez pas si il n'avait pas de médecin traitant fait le 15, appeler le SAMU, vous y trouverez des professionnels, des professionnels compétents qui pourront vous diriger vers le meilleur parcours de soin pour votre enfant, je le redis, qui n'est pas toujours l'hôpital mais qui est le plus souvent le le médecin traitant, je vous invite à aller voir ces professionnels à Bordeaux par exemple ou à Créteil, éventuellement en ce qui concerne la problématique de l'hôpital, je vous rejoins, nous avons des problèmes structurels dans notre hôpital, ils ne sont malheureusement pas nouveau. Un de mes engagements, c'est justement de travailler sur ces problèmes structurels globaux de l'hôpital et pas uniquement bien sûr sur la filière de pédiatrie, c'est ce que porte le PLFSS pour l'année prochaine, dont nous aurons l'occasion je pense de discuter dans les semaines qui viennent, plus librement vous détailler l'ensemble des mesures pour restructurer notre système de santé à l'hôpital public. La parole est maintenant notre collègue Serge mais Rio pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État en charge de la ruralité, mes chers collègues, travailler main dans la main avec les élus ruraux, vous l'avez promis le 19 octobre dans la presse, ce même jour, l'AMF sortait un rapport sur la nécessaire préservation du dispositif des zones de revitalisation rurale, or, sur ce sujet, les élus attendent toujours une main tendue pour l'heure, pas de calendrier, pourquoi tant d'opacité de la clarté, voilà ce qu'exige la ruralité depuis 95 les ZRR sont un facteur essentiel du développement et de l'attractivité de nos territoires, leur fait en décembre 2023 inquiète les élus ce dispositif concerne aujourd'hui près de 14000 communes et un gage 320 millions d'euros, une somme dérisoire au vu des effets positifs observés sur le territoire, implantation d'entreprises de médecins d'acteurs économiques, bref, il a su qu'ont contribué à redonner vie à nombre de nos villages, le rapport sénatorial d'avril 2000 22 et les ruraux salue son efficacité, à l'instar de l'AMF, il vous demande de reconduire un dispositif réformer, prenant en compte les évolutions des territoires en concertation avec leurs élus, revenir à l'échelle des communes et toute une de niveau de classement et toute une série d'autres mesures, bref, le travail, vous avez prémâché emparez vous en posant les fondations d'une nouvelle politique de dynamisation des zones rurales en ces temps troublés pour les collectivités locales, nous devons les accompagner les concertée et leur donner de la visibilité Madame la, à la ministre, quels dispositifs entendez-vous mettre en place pour pallier la disparition des ZRR, quelle place auront les élus dans l'élaboration de ce dispositif. On vous répond : la parole est à madame la secrétaire d'État en charge de la ruralité Madame Dominique Faure, vous avez la parole de Madame la Ministre. Merci, merci, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Serge Méry ou les zones de revitalisation rurale les ZRR ont été créées par la loi d'orientation et d'aménagement. et du développement du territoire le 4 février 95 et je sais le rôle déterminant qu'a je vous le Sénat dans l'adoption de cette loi. Le législateur a souhaité prendre en compte les difficultés spécifiques liés au maintien d'activité en milieu rural, et de façon plus générale soutenir des parties de notre territoire qui sont en déprise démographique économique pour atteindre ce but, les ZRR ont été adossé un régime d'exonération fiscale et sociale aujourd'hui ses 13712 communes qui sont classées en ZRR et qui représentent 16 % de la population française, je suis très attaché à ce dispositif, qui qui prend fin au 31 décembre 2023 et qui reconnaît la fragilité des territoires ruraux, afin de préparer l'avenir, le 1er ministre Jean Castex avait confié une mission parlementaire au sénateur Espagnac et Delcros et aux députés blancs et cette cette prorogation et cette mission parlementaire témoigne de notre attachement commun à ce dispositif, aujourd'hui, il convient de poursuivre le travail que nous avons engagé pour en définir l'avenir depuis mon entrée au gouvernement, et dès le 26 juillet, quelques jours après ma prise de fonction, je répondait à l'invitation du sénateur Delcros de travailler sur cette question le 25 août J. planchait avec le président de l'AMRF et certains membres de son bureau le 8 septembre avec les co-présidente de la commission ruralité de l'AMF cet après-midi même, je reçois officiellement les auteurs de la mission parlementaire avec Christophe Béchu, nous ferons un 1er, travail sur les 14 propositions du rapport, vous le voyez, le gouvernement et donc au travail pour envisager l'avenir des ZRR nous avons confié une mission d'appui avec la DGCL à monsieur François Philizot, inspecteur général et président du conseil d'orientation de l'Observatoire des territoires afin de faire des propositions avec Christophe Béchu à la première ministre au début de l'année 2023 ces propositions se nourriront de travail de large concertation avec le groupe ruralité en cours de constitution à l'Assemblée nationale et je l'espère, avec un groupe ruralité institutionnalisée au Sénat si vous deviez le décider monsieur notre Madame la Ministre, ces concertations seront complétées par des rencontres avec des associations. Salut je. Croyez bien monsieur le sénateur que je vous tiendrai informés de nos travaux, je mettrai toute mon énergie à ce que le gouvernement continue de reconnaître la fragilité des territoires ruraux, vous terminez

donner leur donner aux territoires ruraux, les moyens nécessaires, tant qu'il est encore temps. Monsieur le Ministre, samedi se tenait en Savoie, une conférence de presse destinée à présenter la tribune cosignée par élus, syndicalistes, représentants des associations, élus locaux et parlementaires, nous étions plus de 200 de toutes sensibilités politiques confondues, nous souhaitions rappeler nos engagements pour le chantier ferroviaire du Lyon-Turin et notre choix du scénario grand gabarit pour ses accès à la suite de la consultation que vous avez mené le gouvernement devait prendre une position officielle en début d'année, ce n'est toujours pas fait, je vous rappelle mes courriers restés sans réponse, de plus, en l'absence de décision vous ouvrez une brèche à une minorité d'activistes qui se disent écologistes mais sont contradictoires dans leurs discours, ils cherchent à effrayer nos populations par la désinformation en s'appuyant depuis plus de 30 ans sur les thèmes à la mode du moment roche radioactive amiante y faire et aujourd'hui avec les sécheresses, il pointe les atteintes aux sources d'eau pourtant l'entreprise binationale tels que celui de façon très sérieuse ce sujet en lien avec les élus locaux, c'est par le ferroutage que nous réussirons à diminuer nos émissions carbonées et à améliorer la qualité de l'air dans nos vallées, la ligne historique n'en a pas la capacité, et nous devons en parallèle libérer des sillons pour les transports voyageurs du quotidien la légitimité démocratique à faire des choix qui engagent l'avenir de nos enfants appartient bien aux élus et non à une poignée de militants opposés au projet, monsieur le Ministre : Ne vous laissez pas impressionner prenait les décisions attendues, la question n'est plus d'être pour ou contre ce tunnel, il s'agit d'en déterminer ses accès et d'en assurer leur financement aussi mes questions sont simples: quand comptez-vous confirmer officiellement le scénario retenu, d'autre part, l'Union européenne a annoncé 50 % de financement pour les accès, vous n'avez pas postulé à son appel à projets opérations ferroviaires, alors que le percement du tunnel est en cours, quand le ferez-vous. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des transports Monsieur bonne. je partage pour être très clair avec vous, l'engagement et l'intérêt incontestable de ce projet, il est important sur le plan écologique, vous l'avez rappelé pour le développement du ferroviaire et du fret ferroviaire, en particulier, il est essentiel pour les mêmes raisons, sur le plan économique et c'est un grand projet européen que nous devons faire avancer, il a été d'ailleurs confirmé au plus haut niveau dans le traité d'amitié entre la France et l'Italie, il y a moins d'un an, les concertations ont été engagés, selon un calendrier que vous connaissez, qui est transparent par le préfet de région, le préfet Pascal maillot il y a eu concertation avec les élus, toutes les collectivités qui peuvent être amenées à financer la question des accès et ce travail s'est terminé au début de l'année 2022 dès que je suis arrivée, j'en ai pris l'engagement devant le Parlement dès le mois de juillet, j'ai repris le travail de concertation pour que nous passions maintenant la partie concrète et financière, je me suis rendu comme je l'avais indiqué à Lyon dès le mois de septembre pour échanger avec l'ensemble des collectivités financeurs, j'ai constaté, comme vous l'avez rappelé que le scénario qui avait la nette préférence de l'immense majorité des collectivités, c'était ce scénario pour les accès dit grand gabarit et et maintenant, j'ai demandé qu'il y a une concertation et j'ai mandaté le préfet à cette fin, d'ici le début de l'année prochaine pour qu'en face de cette ambition ferroviaire il y a une ambition budgétaire car le scénario grand gabarit est aussi le le scénario grand gabarit est aussi le scénario le plus coûteux, et donc si les collectivités sont prêtes à s'engager, nous le serons aussi il faut que maintenant chacun dit ce qu'il est prêt à mettre concrètement de manière sonnante et trébuchante, sur la table, nous sommes prêts à nous engager pour se faire et à mobiliser aussi les financements européens sur la section transfrontalière dans le PLF 2023 qui est bientôt soumis à votre débat, des crédits sont là intégralement toute la programmation respecter, j'ai eu encore hier un entretien avec la Commission européenne pour que les financements sur cette section transfrontalière soit rapidement mobilisés, il n'y a aucun désengagement à cet égard et quand le scénario sur les accès sera arrêtée sur le plan ferroviaire et budgétaire nous postuleront évidemment financements européens et, comme vous l'avez rappelé en effet : l'Union européenne nous a indiqué qu'elle était prête à mobiliser 50 pour 100 des financements jusqu'à 50 % des financements sur cet accès et l'État sera au rendez-vous, mais il faut que tout le monde soit au rendez-vous, les collectivités, l'État, j'ai pris cet engagement au nom de l'État au mois de septembre, nous attendons maintenant la concertation financière d'ici le début de l'année, je crois que cet engagement a été pris au mois de juillet, il est tenu. Merci, c'est d'ailleurs dans l'article 10. De du projet de traité que vous allez examiner mes chers collègues, à partir de 16 heures 30 et donc c'est confirmé votre votre nous permettra d'examiner ce point. Et je me permets de le souligner, la parole est maintenant notre collègue François Bonneau pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la transition énergétique, la crise de l'énergie que nous connaissons et sans précédent, si la situation semble revenir à la normale sur le front des carburants, nous devons nous préparer à des coupures d'électricité et de gaz, sans être certaine ces coupures sont possibles : la guerre en Ukraine et ses effets atroce sur sa population étant malheureusement le révélateur d'une situation qui se dégrader depuis plusieurs années, faute d'anticipation pour l'électricité, la moitié des réacteurs nucléaires est encore à l'arrêt et EDF ne cesse de différer leur remise en service, à cela s'ajoutent les grèves dans les centrales qui réduisent encore un peu plus nos capacités de production et l'effort de maintenance, les énergies renouvelables, bien qu'importantes, son nom pilotable en absence de vent et le soleil et nucléaire, ce sont les centrales à gaz qui prendront le relais, nous approchons de la période hivernale et certains spécialistes nous annoncent qu'ils pourraient être rigoureux, s'agissant du gaz nos réserves sont pleines, mais elle ne représente que les 2 tiers de la consommation hivernale des PME et des particuliers, les entreprises Gazou intensives ont déjà été prévenus qu'elle pourrait avoir à subir des coupures préjudiciable à leur activité, les Français sont prêts à faire des efforts, mais accepteront mal de ne pas être prévenu et alerté à temps, ma question est donc : comment allez-vous procéder vis-à-vis des entreprises pour les inciter à s'arrêter avec quel délai et pour combien de temps. Comment allez-vous procéder à l'égard des particuliers, des collectivités, des établissements scolaires à à quels horaires selon quel délai comment organiser ces coupures pour les situations particulières médicale ou sociale qui utilisation ferez-vous des compteurs Linky a a bien nommer les choses ont contribué à régler les problèmes du pays. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Bono, vous avez raison de mentionner cette plus grave crise énergétique que nous connaissons depuis les années 70 avec le quasi-arrêt des livraisons en Europe du gaz russe, de quoi par le ton de 40 % du gaz qui approvisionner l'Europe et qui aujourd'hui crée un stress sur notre système énergétique, ce n'est pas propre à la France, c'est propre à l'Europe et nous agissons ensemble en solidarité nous avons également à faire face à une moindre production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique du fait des sécheresses, que nous avons connu cet été et pour le nucléaire, vous l'avez mentionné de souci de maintenance sur lequel nous agissons

en France, mais également dans toute l'Europe, à l'initiative de la France, je le rappelle, l'augmentation de nos capacités d'approvisionnement en gaz naturel, les stocks sont remplis mais les terminaux continue à acheminer du gaz à pleine capacité, l'augmentation de la puissance de certains barrages hydrauliques, la préservation de nos capacités de production cet été pour les réserver à l'hiver, je ne vais pas mentionné toutes les décisions que nous avons prises pour préserver cet hiver vous mentionnez la situation d'EDF et je veux saluer ici l'accord qui a été trouvé au niveau de l'entreprise d'EDF et la reprise du travail, qui s'est fait ce week-end pour précisément faire en sorte que, on continue à agir sur les maths ça remettre en état nos centrales nucléaires pour qu'elle puisse produire cet hiver et cela a été fait en grande responsabilité par les organisations syndicales et par la direction d'EDF enfin quelles sont les actions, vous le savez, RTE, qui est notre expert en la matière, mentionne des risques très limité de difficultés cet hiver si l'hiver est normal en termes de température et donc par rapport à la Syrie très limité, nous agissons, nous avons interruptibilité effacement sécurisation des interconnexions, et s'agissant du scénario ultime de coupure là encore un plan est activé et on ne parle que de 2 heures d'interruption par jour en matière d'électricité, je dirais pas plus loin, temps est largement dépassé. Oui, madame la Ministre, permettez-moi d'insister sur les coupures de gaz qui pourraient toucher les entreprises notamment cette s'agissant de la durée de ces coupures, il faudra que ce soit vu en amont et en concertation, parce que ça peut avoir des conséquences très graves pour vingt entreprises ainsi. nos prochaines questions d'actualité, auront lieu le mercredi de devant ma 15 heures je vais maintenant suspende la séance, elle sera reprise à 16 heures 30 pour l'examen de conventions internationales, la séance est suspendue.

La séance est reprise en application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de ordinaire prises pour son application, la commission des affaires économiques, a émis lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable 26 voix pour, 19 voix contre à la nomination de Monsieur Luc Rémont aux fonctions de président directeur général d'Électricité de France. Assemble Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement, l'ordre du jour appelle l'examen de 4 projets de loi tendant Ohrid d'autoriser la ratification l'approbation de conventions internationales pour ces 4 projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifiée, je vais donc les maîtres successivement aux voix je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives, la commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte qui est pour, qui est contre qui s'abstient le projet et donc adopté je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidentale et de la cour régionale sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien lancé la commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte qui est pour, qui est contre un qui s'abstient le projet doit être adopté je mais aux voit le texte adopté par la commission sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après un engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatifs au statut et aux activités de la Banque des règlements internationaux en France et de l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux, la commission des Affaires étrangères est favorable, l'adoption de ce texte Qui est contre qui s'abstient-il être adopté définitivement je mais on voit le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, la commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte qui, pour

du traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée dans la discussion générale, la parole est est à Madame Laurence Boone, secrétaire d'État chargé de l'Europe. mène, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, je suis donc aujourd'hui à votre disposition pour débattre avec vous, du projet de loi visant à ratifier le traité pour une coopération bilatérale renforcée entre la France et l'Italie 10 traité du Quirinal, comme vous le savez, il a été signé, entre nos 2 pays le 26 novembre 2021 à Rome et ce projet de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale le 28 juillet dernier. Le traité du Quirinal et le 1er traité de portée générale, et de cette ampleur avec l'Italie, il aura pour vocation de façonner pendant les prochaines décennies, l'histoire de la relation franco-italienne. Le choix du palais présidentiel italien sur la colline du Quirinal pour accueillir la cérémonie de signature, a ainsi témoigné du caractère exceptionnel et historique de cet événement auquel ont assisté les plus hautes autorités de nos 2 pays. Entre-temps, un nouveau gouvernement italien a pris ses fonctions le 22 octobre sous la présidence de madame Meloni c'est une nouvelle phase pour l'Italie et la nouvelle présidente du conseil a pu s'en entretenir avec le président de la république dimanche dernier à Rome. C'est sans doute une phase où des différentes politiques trouveront à s'exprimer entre nos gouvernements comme c'est légitime entre 2 démocratie. Et c'est aussi une phase et je veux le dire ici, dans laquelle la France reste convaincu que nous devons poursuivre l'ambition du traité du Quirinal. Qui est celle d'exploiter davantage l'immense potentiel de nos relations. Celle-ci s'appuie sur une amitié de longue date, riche d'échanges entre nos 2 États mais aussi et surtout entre nos 2 peuples nous, société civile, nos intellectuels, nos économies qui communiquent et interagissent naturellement depuis des siècles et parfois au sein d'un même bassin de vie. Je. Donc quel est notre objectif avec le traité du Quirinal ces 2 structurer encore davantage nos échanges et nos coopérations grâce à un cadre institutionnel formalisé à tous les niveaux de coopération. Depuis la signature de ce traité ces échanges et ces coopérations ont déjà commencé à se structurer et à se renforcer au niveau national, bien sûr, mais aussi au niveau des régions des communes de la société civile et des acteurs économiques. Cette habitude de travail doit nous permettent d'approfondir nos coopérations sur les sujets d'intérêt commun. Elle vise aussi à stabiliser dans la durée, une relation qui a parfois connu, vous le savez, Des hauts et des bas, il a ancré dans le temps long, au service de nos peuples et au service de l'Europe. Le traité du Quirinal se veut profondément européen dans ses valeurs et dans ses objectifs. Et il nous rappelle combien les convergences entre la France et l'Italie ont constitué l'un des ciments du projet européen, il traduit aussi l'ambition de travailler ensemble, face aux défis considérables auxquels est confrontée l'Union Européenne aujourd'hui. L'Italie est évidemment un partenaire indispensable pour porter l'agenda de souveraineté et d'autonomie stratégique de l'Union européenne pour préserver l'unité européenne et pour développer ou plutôt continuer de développer une réponse commune face à la guerre en Ukraine. C'est pourquoi les coopérations bilatérales qui sont prévues par le traité, ont elles aussi une dimension européenne, puisque le but et qu'elle contribue à renforcer notre union, y compris par une meilleure intégration de nos territoires. Mesdames et messieurs les sénateurs, je souhaiterais à présent revenir sur quelques dispositions clés du traité. D'abord le traité fixe l'objectif d'un approfondissement de nos coopérations en matière de défense évidemment la pertinence de cette co-de ces coopérations croit davantage encore avec le retour de la guerre, sur notre continent, il souligne également la solidarité qui lie nos 2 pays en cas d'agression de nos territoires respectifs et comme vous le savez, cette disposition est conforme aux engagements internationaux auxquels nous avons souscrit notamment la charte du traité de l'Atlantique nord, et de pardon, mais néanmoins c'est un symbole fort, à fortiori à nouveau dans le contexte international dégradé que nous connaissons et qui demande plus que jamais à renforcer notre unité. Deuxièmement. Le traité fait de la Méditerranée dès son préambule, un espace de coopération privilégiée. Cet espace stratégique et la Méditerranée pour nos 2 pays doit évidemment être au coeur de la coordination franco- italienne sur de nombreux plans qu'il s'agisse de politique de voisinage, de développement et d'économie bleue de sécurité, d'environnement, il doit aussi faire l'objet de toute notre attention, dans le cadre de notre coopération bilatérale autour de la gestion de notre frontière maritime commune. Troisièmement, et c'est presque le dernièrement construisant sur une relation économiques déjà intenses, le traité prévoit que la France et l'Italie favoriseront les rapprochements équilibré entre les acteurs économiques. Cette proximité doit permettre une meilleure connaissance réciproque entre les entreprises françaises et italiennes et favoriser la présence et le développement mutuellement bénéfique des industries de nos 2 pays dans de nombreux secteurs, mais par exemple, l'autonomie stratégique européenne, le numérique, la transition écologique ou encore l'industrie spatiale. Quatrièmement, le développement d'une coopération transfrontalière transversale, un autre objectif 1 % du traité doit permettre la réalisation de projets concrets au bénéfice des habitants des régions frontalières, ces projets peuvent concerner les enjeux de mobilité de secours de développement économique et également de protection de l'environnement. Un comité de coopération frontalière qui était inspirée du modèle franco-allemand et qui associe les parlementaires est instituée par ce texte. Il permettra, il a été très utile dans le cas des frontières avec l'Allemagne, de porter des projets conjoints en levant les obstacles souvent réglementaire, mais pas seulement réglementaire qui sont liés à la frontière. Enfin, il y a un focus spécial sur le rapprochement de nos jeunes et c'est vraiment un axe fort de ce traité et nous allons construire une véritable stratégie pour favoriser des Liens durables entre les jeunes Français et les jeunes. Ainsi, Ainsi, un service civique franco-italien sera mis en place avec un objectif de 150 volontaires qui effectueront chaque année une mobilité entre la France et l'Italie, et bien sûr il y aura la mobilité ou des mobilités, je devrais dire des élèves des apprentis et des étudiants. Voilà, je ne vais pas évoquer devant vous, l'ensemble des dispositions de ce traité, extrêmement riche, car cela nécessiterait beaucoup plus que quelques minutes, ce que je voudrais simplement vous redire, c'est que ce traité, si vous le ratifier sera structurant pour l'avenir de notre relation de long terme avec l'Italie et que nous nous attacherons à sa pleine mise en oeuvre. Vous rappeler aussi que c'est un enjeu qui est particulièrement important pour les populations vivant à la frontière. pour finir je je souhaiterais terminer mon intervention, on a en évoquant un aspect central de la relation institutionnelle franco-italienne, celui de la diplomatie parlementaire, il est indispensable que nos 2 parlements soient pleinement impliqués dans le dialogue franco-italien et à cet égard je sais toute l'implication des présidents Jean-François Rapin et Hervé Marseille, cette assemblée a déjà avancé sur la structuration de ses relations avec le Parlement italien et je m'en réjouis, je tiens également à saluer les échanges ancien entre groupes parlementaires d'amitié, de part et d'autre des Alpes, je suis convaincu qu'ils seront à nouveau très utile sous cette législature voici monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les principaux éléments que je souhaitais porter à votre connaissance sur ce traité de coopération bilatérale renforcée entre la France et l'Italie, je vous remercie.

Madame la présidente, madame la ministre, madame l'ambassadrice d'Italie en France. Nous, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi autorisant la ratification du traité. La République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée, mieux connu sous le nom du traité de Quirinal non du palais présidentiel, où il a été signé le 26 novembre 2021, par le président de la République française, Monsieur, Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Monsieur Mario Draghi, qui, en présence du président italien Sergio Mattarella ce texte. A été adopté en commission lors de sa réunion du 27 septembre le groupe écologiste solidarité Thierry. A souhaité le retour à la procédure normale afin qu'il soit débattu dans cette convention de partenariat, ce que j'approuve totalement, toutefois je tiens à. Voulez que nous ne pouvons pas amender ce projet de loi qui soit, qui sera soit adopté soit. Rejeté par notre assemblée l'actualité politique italienne apporte un éclairage nouveau sur nos relations bilatérales. Qui ont déjà connu Des hauts et des bas ces dernières années au printemps 2018. L'arrivée au pouvoir de l'alliance entre la Ligue, parti d'extrême droite et le Mouvement 5 étoiles a fait prospérer les narratif anti-élites et anti-européen, voire anti-français le summum de la crise est atteint. Lorsqu'en janvier 2019 le vice-. Président du Conseil, monsieur Di Meh di Maio nous Mouvement 5 étoiles apporte son appui au moment des gilets jaunes, l'ambassadeur français Christian Masset a été. En France, le 7 février 2019 ce n'était pas arrivé depuis 1940. Lorsque Mussolini avait déclaré la guerre en France encore récemment la vie de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, rendu le 29 juin 2022 défavorables à la mise à. Exécution des demandes d'extradition de 10 anciens militants d'extrême gauche pour faits de terrorisme ah. Thomas ému l'opinion publique italienne, les propos tenus par le président de la République française et l'annonce d'un pourvoi en cassation par le parquet, ont eu un fort effet d'apaisement en Italie. à quelques jours seulement de la ratification du président. Prêté par le Sénat italien à l'été 2019 la constitution d'une nouvelle coalition composée du Mouvement 5 étoiles et du Parti démocrate, puis l'arrivée de Mario Draghi à la présidence. C'est du Conseil en février 2000 21 ans, permis de relancer le processus. ASUS du traité de Quirinal les excellentes collaborations bilatérales entre la France et l'Italie, soutenue par différents secteurs de la société civile ont également contribué au rapprochement. Aboutissant à la signature du traité le 26 novembre 2021 les domaines de coopération prévue par le traité. Et son parti qui leur nom étendu concerne les affaires étrangères, la sécurité, la défense, les affaires européennes, les politiques migratoires. Justice et affaires intérieures, la coopération économique, industrielle et numérique, les droits sociaux. Le développement durable, l'espace, l'enseignement et la recherche, la culture et la jeunesse, et enfin la coopération transfrontalière, les objectifs de coopération. Sans préciser et décliner de manière plus opérationnel dans une feuille de route. Qui est révisable chaque année en fonction de l'évolution des priorités et de l'environnement international et européen, la première version de cette feuille de route a été signé en même temps que le traité plusieurs mécanismes de consultation et de coopération. Sont prévues par le traité, enfin de développer une culture administrative commune et des habitudes de. Consultation qui favoriseront l'émergence de réflexe franco-italien ce rapprochement sera favorisé. Par les formats de consultation régulier, inscrit dans le dans le traité pour tous les domaines, la mise en oeuvre du traité est assurée par un comité stratégique. Paritaire au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, le traité prévoit un certain nombre d'espace d'échange au niveau interministériel et administratif ainsi. Par exemple hein gouvernemental, il est prévu la relance du conseil franco-italien de défense. Et de sécurité, un forum de concertation économique des réunions bilatérales annuelles pour différents ministres un dialogue sur les transports de plus chaque trimestre un membre du gouvernement de l'un des 2 États doivent prendre part au conseil des ministres de l'autre État. Au niveau administratif, plusieurs l'instance de concertation thématiques sont prévenus sont prévus comme en maths. Terre d'immigration et asile ou de sécurité intérieure ainsi que l'échange de fonctionnaires pour les sociétés civiles, le texte prévoit un autre. Notamment la création d'un conseil franco-italien de la jeunesse et la mise en place d'un service civique franco-italien ce réflexe. Franco-italien trouvera également une traduction au niveau européen, le traité prévoit dans son article 3 que les 2 États présenteront des. Position commune au niveau européen, notamment sur le recours à la majorité qualifiée étendu ou l'adoption de. Voilà le règle budgétaire la feuille de route, fait d'ailleurs expressément mention de la révision du pacte de stabilité, le sujet de la réforme de la politique européenne migratoire et d'asile, a fait l'objet de négociations plus soutenu. Un compromis a été trouvé en faisant référence à une réforme, hein. Frondeur et une mise en oeuvre efficace de la politique migratoire et d'asile européenne il faut souligner que le traité prévoit le volet parlementaire dans son préambule, le texte reconnaît l'importance et la vitalité de la. Coopération entre leurs parlements respectifs et le rôle de la que la diplomatie parlementaire joue dans les Liens entre leur pays et souhaitent la renforcer. à travers des formes de coopération permanente, notamment entre leurs commissions respectives, l'Assemblée nationale et la Chambre des députés ont d'ailleurs déjà conclu un protocole de coopération le 29 novembre 2021, la commission des Affaires étrangères. De la Défense et des forces armées a pour sa part effectuer un déplacement en Italie du 1er au 4. Décembre 2021 menée par notre président, Christian Cambon au cours duquel la con. Fusion d'un accord de coopération avec le Sénat italien a été évoquée, il faut souligner. Traité comme celui du Quirinal est très rare en Europe, il s'agit seulement du second traité signés par la France après celui de l'Élysée, paraphé en 1963 complété par celui d'Aix-la-Chapelle en 2019 avec l'Allemagne, le traité du Quirinal a été ratifiée en Italie. Par la Chambre des députés, le 25 mai et par le Sénat le 5 juillet à chaque fois à une très grande majorité au Sénat, seuls les sénateurs d'opposition. Fratelli d'Italia et quelques noms inscrits anti-européen dissidents du Mouvement 5 étoiles ont voté contre 28 voix et se sont abstenus, 5 en France, l'Assemblée nationale s'est prononcée à l'unanimité. C'est des suffrages exprimés pour sa ratification le 20 juillet 2022. Le Sénat, et donc la dernière chambre à être saisi du projet de loi la coïncidence entre l'examen par le Sénat du présent projet de loi avec elle investi. Dur de Giorgia Giorgia Meloni comme présidente du conseil fait que nous devons nous interroger. Sur la volonté de cette dernière à mettre en oeuvre le traité de Quirinal, en effet, on se souvient que ce sont majoritairement les parlementaires de son parti. Fratelli d'Italia, qui ont voté contre la ratification du traité leur principal argument était d'avoir tenu dans l'ignorance du. Texte et qu'en tant que parti d'opposition, il ne pouvait signer un chèque en blanc au gouvernement plus implicitement il considérait le traité comme. Cependant avant tout les intérêts français. Dans une récente interview. Georgia Meloni, ne pas être con, convaincu par l'idée de poursuivre l'intégration. Au moyen de traités bilatéraux mais que maintenant que le traité est en vigueur et nous donne un cadre, il appartient au gouvernement et aux hommes politiques, de lui donner encore tenue. On peut constater qu'à l'approche du pouvoir Giorgia ah Meloni, hein, mais de l'eau dans son vin le programme. De la de sa coalition, prévoyez le respect des alliances internationales désengagement contre l'Alliance Atlantique et du soutien à l'Ukraine face à l'invasion de la Fédération russe été la seule. à soutenir, sans ambiguïté, le gouvernement Draghi pour le plan international sur l'envoi d'armes à l'Ukraine sur l'Europe. Elle a exprimé son souhait est une Europe plus stratégique plus géopolitique au sein de laquelle l'Italie devra prendre toute sa place, les récents propos tenus par Silvio Berlin. Sur sa proximité avec ma Didine Poutine ont pu choquer, mais les élections des présidents des Chambres elle est. Ministériel ont démontré que la corrélation est par elle et que le fondateur de Força Italia ne passe sans doute pas autant autant qu'il affirme enfin si des positions différentes sur un certain nombre de sujets bon certainement voir le jour. Ne faut-il pas capitaliser sur ce qui pourrait nous rapprocher la mise. Ah en Oeuvres du traité du Quirinal, notamment dans le secteur de l'armement et de l'espace pour, à ce titre, jouer un rôle d'un test pour nos relations bilatérales, la visite d'Emmanuel. à Rome, le week-end dernier à l'occasion du Forum pour la paix, Marc, cette volonté de maintenir le dialogue et son respect pour le choix démocratique des Italiens, pariant sur la victoire du. Réalisme sur les néologie je préconise l'adoption de ce projet de loi autorisant la ratification du traité du Quirinal sur lequel je vous le rappelle, le Sénat et la dernière des quatre chambres à se prononcer, merci. Merci dans Merci dans la discussion générale, la parole est au président Hervé Marseille pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant de commencer mon propos, permettez-moi de saluer son excellence Madame et Manuela d'Alessandro, nouvelle ambassadrice d'Italie en France qui nous fait l'honneur de sa présence dans cet hémicycle à la tribune présidentielle merci excellence. Connu sous Connu sous le nom de traité du Quirinal, le traité de coopération bilatérale renforcée entre l'Italie et la France a fait l'objet de nombreuses et longues négociations après une crise diplomatique et a une crise sanitaire, il a finalement été conclu le 26 novembre dernier au palais du Quirinal ce traité vient sceller une relation dense privilégier une longue amitié entre nos 2 pays, comme vous le savez, l'Italie et la France font partie des pays fondateurs de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis de la communauté européenne économique depuis l'origine, l'Europe, on le voit bien, c'est aussi l'énergie, le traité de Rome signé en 1957 dans la capitale italienne et d'ailleurs, une reconnaissance du rôle essentiel joué par l'Italie dans la construction du projet européen, nos échanges politiques avec l'Italie existe depuis longtemps, et des sommets bilatéraux ont été organisés sur différents sujets, pour autant, le manque de cadres et d'habitude dans les relations diplomatiques pour pardon politique entre nos 2 États expose trop dangereusement les relations bilatérales aux variations de majorité tant en Italie qu'en France la ratification permettra à nos représentants respectifs d'exposer sur la scène internationale et européenne des positions mieux accordé et donc plus influentes le traité du Quirinal s'inscrit dans l'esprit du traité de l'Élysée de 1963 celui-ci avait posé les jalons du couple franco-allemand et donner une base solide à une coopération régulière, il a aussi impulser un dialogue systématique entre l'Allemagne et la France, la France et l'Italie ont 515 kilomètres de frontières communes et partage à la fois des espaces naturels des infrastructures et des bassins de vie, les enjeux de cet espace frontalier sont donc multiples, sécurité, environnement économique ou encore liés au transport de voyageurs et de marchandises, le traité du Quirinal à un objectif simple organiser la relation bilatérale en lui donnant un cadre et des orientations stratégiques qui permettront de l'inscrire dans la durée les négociations entamées depuis 2018 avaient alors montré la grande proximité de nos 2 gouvernements et notre convergence sur de nombreux objectifs, notamment européens, je souhaite rappeler ici quelques propositions essentielles et concrète que promu le traité une politique étrangère ayant vocation à stabiliser et préserver la mer Méditerranée occidentale et orientale, ainsi qu'une meilleure concertation de nos pays pour la défense de position communes au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, une politique de défense qui instaure une collaboration stratégique étroites et de haut niveau avec une assistance mutuelle en cas d'agression sur le territoire de l'un d'entre eux, une politique de sécurité à travers la création d'une unité opérationnelle franco-italienne dont l'ambition est de mieux coordonner les actions contre les réseaux d'immigration clandestine, la criminalité et la corruption et la fraude s'agissant de l'immigration, je vous rappelle combien dans ce domaine, l'Italie a souvent été abandonnées à elles-mêmes et combien il faut accompagner les efforts dans ce sens, une politique agricole qui privilégie et protège la qualité des produits, les AOP, les IGP, l'instauration d'un service civil commun pour les jeunes, il prévoit l'invitation régulière de ministres au conseil des ministres respectifs, sur le modèle du traité d'Aix-la-Chapelle le traité assure également un volet parlementaire en reconnaissant l'importance de la coopération entre nos parlements respectifs la Ministre de l'avoir souligné dans votre propos ainsi que mon collègue boucher le 25 septembre dernier les Italiens ont choisi de placer à la tête de leur pays, madame Meloni madame Meloni, avait alors déclaré à propos du traité du Quirinal, que c'était un acte qui n'était pas démocratique car le Parlement italien n'avait pas été consulté et qu'il servait avant tout les intérêts français, elle avait même dénoncé un impérialisme français et lors de l'examen de la ratification au Sénat italien le rapporteur, la cité le parti Fratelli d'Italia et ses alliés ont voté contre la ratification du traité ou se sont abstenus, on considérera qu'il s'agit de péripéties de campagne, même si ils sont préoccupants, cette position peut faire naître des doutes sur la mise en oeuvre de l'application du traité pour autant des signes encourageants et des clarifications ont été donnés depuis ainsi hier, lors de sa déclaration de politique générale, la présidente du Conseil italien a rappelé à dessein que l'Italie faisait pleinement partie de l'Europe et qu'elle souhaitait une intégration européenne plus efficace Madame la Ministre, le président de la République a pu rencontrer madame Meloni lors de son déplacement en Italie le week-end dernier et je considère que c'est une bonne chose, le sujet a été bien évoqué dans leurs échanges, j'espère que vous pourrez nous apporter des éclaircissements dans dans ce domaine est-ce que la mise en oeuvre du traité, hé bien à l'ordre du jour des agendas politiques respectifs, peut-être pourrez-vous nous éclairer sur cet aspect des choses, vous avez compris que le groupe Union centriste appelle de ses voeux toute action en ce sens à l'heure où les équilibres mondiaux sont bouleversés et que la guerre a fait son retour sur le sol européen, il est plus que nécessaire de sceller durablement entre la France et l'Italie, une coopération historique et des ambitions communes l'impulsion décisive du gouvernement de Monsieur Draghi et le précieux concours du président Mattarella ont abouti au traité du Quirinal qui ne doit pas être ralentie pour le bien de l'Europe à laquelle les 2 pays travaillent depuis longtemps, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe Union centriste bien sûr votera favorablement à la ratification de ce traité et je vous en remercie. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous devons approuver aujourd'hui la ratification du traité de coopération bilatérale renforcée entre la France et l'Italie, il y a quelques mois, cette étape, on n'aurait pas suscité beaucoup de commentaires, bien que tumultueuse, vers la fin de la dernière décennie, nos relations avec les avec l'Italie, ont connu depuis une embellie, c'est d'ailleurs dans ce contexte d'apaisement diplomatique entre Paris et Rome, que le traité de lui dit du Quirinal a dû être signé, a pu être signé sans ombrage le 26 novembre 2021, oui mais voilà, les récentes élections législatives en Italie ont porté au pouvoir, Georgia Meloni une situation politique chargé d'inquiétude qui disons le justifie à elle seule notre débat d'aujourd'hui, le parti d'extrême droite Fratelli l'Italien de la première ministre et de la prétendue admiration de celle aussi pour Mussolini sont ont en effet de quoi nous interroger, j'ajouterai qu'au sein de son équipe gouvernementale entre les propos pro-poutinien de certains et les discours conservateur des autres, il est clair que pèse un risque sur les valeurs auxquelles la France est attachée, pour autant, ne doit-on pas dissocier le traité, un engagement de long terme entre la France et l'Italie de la nouvelle donne politique italienne par nature conjoncturelle, les dirigeants de tâches et les traiter dur parce qu'il engage, nos 2 pays sur la voie de la coopération étroite dans de nombreux domaines, cet accord n'est-il pas au fond un des moyens de maintenir l'Italie dans les clous de la démocratie, la multiplication des échanges dans ton nos administrations, nos économies et nos territoires en particulier frontaliers, l'article 9 du traité qui place à la jeunesse au coeur de la relation franco-italienne sur le plan de la défense, l'engagement de renforcer les coopérations internes de capacité hein et opérationnel spatial et industriel. Tous ces vols et devrait permettre de conforter notre amitié avec l'Italie, un pays avec lequel, rappelons-le, nous avons la culture latine un partage ce traité, c'est aussi un levier pour une vision commune européenne, comme le rappelle l'article 3 je cite les 2 États oeuvrent ensemble pour une Europe démocratique unie et souveraine et pour le développement de l'autonomie stratégique européenne à à cet égard la première ministre italienne et de donner des gages à Bruxelles en rappelant hier devant ses députés que l'Italie faisait pleinement partie de l'Europe et de l'OTAN, on va juger un peu sur les actes pour reprendre la formule employée par l'Élysée dimanche dernier en effet, nous attendons de voir, mais gageons qu'avec une dépendance économique sur le plan de relance européen post-pandémie de près de 200 milliards d'euros Rome n'a guère d'intérêt à s'éloigner de l'Europe, en retour, il est de la responsabilité de l'Union européenne d'appréhender encore davantage les défis qui parfois mettent l'oeuvre les prêts à l'épreuve, je pense, en effet, à la question migratoire que les pays européens, bordé par la Méditerranée doivent gérer en première ligne le traité bilatéral into la France et l'Italie qui nous occupe aujourd'hui inclut ce sujet et c'est une bonne chose de surcroît si notre pays arrivent à imposer ses valeurs qui sont les siennes, mes chers collègues, ce traité la chance de pouvoir au moins sur le papier un approfondissement de la coopération franco-italienne quant à son application, il est vrai que ceux qui dirigent l'Italie aujourd'hui ne l'ont pas votée lorsqu'il était dans l'opposition, il nous faudra donc être vigilant en attendant il conviendra, si j'ose dire, de tirer vers le haut et d'autoriser la signature de ce traité, approuvé à l'unanimité par nos collègues députés enfin concernant notre confiance au peuple italien car il nous faut garder à l'esprit leurs bonnes intentions originelles et se souvenir aussi un signe d'espoir, d'où vient le champ Bellaciao c'est pourquoi mon groupe approuvera ce projet de loi, je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a peu de nations dans le monde, dont la France peut dire sans emphase excessive, hein, qu'elles sont des nations soeurs l'Italie sans conteste en fait partie, au fil du temps nos relations ont naturellement connu bien des vicissitudes et nos contacts ont été aussi fructueux que tumultueux comment en 20 siècles d'histoire partagée pourrait-il en être autrement face à la richesse de notre passé, comment dresser un inventaire exhaustif des influences que chaque pays que chaque société a eu sur l'autre serait un exercice sans doute impossible la profondeur des Liens qui nous unissent, hein, se retrouve d'ailleurs jusque dans le palais où nous siégeons qui fut construit dans un Style italien pour reine de France venus d'Italie, retenons simplement que si tout au long de l'histoire des guerres ont pu nous opposer que des différents ont pu nous éloigner la culture nous a toujours rapproché, elle est le terreau d'une relation qui trouve ses moteurs dans une géographie commune dans des Liens économiques profonds et dans une nécessité de répondre ensemble aux défis contemporains, ainsi nous avons en partage plus de 500 kilomètres de frontière alpine, de même qu'une partie de la mer Méditerranée, nous y sommes confrontés aux mêmes enjeux environnementaux migratoire ou stratégique avec 82 milliards d'euros d'échanges en 2019 la France et l'Italie sont l'un pour l'autre des partenaires commerciaux de tout 1er plan jusqu'à présent, ce rapport évident, naturel que nous entretenons avec nos voisins transalpins ne se traduisait par aucun traité d'amitié ou de coopération globale, le texte qui nous est soumis aujourd'hui vient combler ce manque, il sanctuarise en quelque sorte notre relation, il la structure la valorise avec en filigrane l'ambition de la hisser au niveau de celles que nous entretenons avec l'Allemagne, nos 2 pays, ainsi que l'Union européenne qu'ils ont contribué à fonder ont naturellement tout à y gagner, bien sûr, nous sommes appelés à en autoriser la ratification au lendemain des élections du 25 septembre qui ont vu les citoyens italiens placé en tête de leurs suffrages, une coalition qui suscite interrogations parfois inquiétude toutefois, permettez-moi de souligner que le peuple italien s'est exprimée souverainement et que son choix doit évidemment être respectée, gardons-nous d'utiliser l'examen du traité du Quirinal comme une occasion d'adresser un message, voire une sanction aux électeurs italiens ou au gouvernement, qu'ils ont choisi et qui vient à peine d'entrer en fonction, d'autant que ce texte réaffirme des valeurs essentielles et qui n'a pas en outre vocation à créer des obligations réciproques, il a pour ambition de proposer une matrice afin de développer un réflexe franco-italien afin de renforcer par les échanges, la compréhension réciproque de nos sociétés et la coopération entre nos institutions, mais c'est bien au gouvernement actuel ou futur aux administrations, collectivités aux sociétés civiles des 2 côtés des Alpes à qu'il appartiendra de faire vivre ou pas le cadre posé par ce traité, celui-ci est appelé se déployer largement, Affaires étrangères, sécurité, défense migration économie enseignement : culture, coopération transfrontalière dans tous ces domaines, la France et l'Italie ont des choses à se dire ah s'apporter mutuellement et apporter à l'Union européenne dans son ensemble, je pense en particulier aux aux dispositions concernant la sécurité et la défense, nul besoin de rappeler dans le contexte actuel dont nous débattrons encore ce soir, qu'il s'agit d'un Champ fondamental pour ne pas dire existentielle, nous faisons face à de nombreux défis à de nouvelles crises dans le bassin méditerranéen, cette situation cette période d'instabilité où les enjeux sont considérables, traduisent l'exigence et la nécessité du renforcement de notre coopération pour la sécurité de l'Europe, nous bénéficions de convergence réelle en particulier ce souci constant de la Méditerranée et de tout ce qui impacte la stabilité de ses rives cette dimension figure d'ailleurs en bonne place au sein du traité mais nous pourrions encore. Procès une vision stratégique qui ne sont pas toujours synchrone à titre d'exemple, si en Italie aussi la réflexion sur l'autonomie stratégique progresse, j'ai pu constater lors d'un déplacement à Rome en fin d'année dernière, que nous ne mettions pas forcément les mêmes choses derrière un même concept nos collaborations industrielles intense mais limitée à une poignée de secteurs ainsi que notre coopération opérationnelle mériterait également d'être étouffée, je me réjouis donc. Que le traité sa feuille de route institut si un dialogue stratégique soutenu et qu'ils mettent l'accent sur les synergies capacitaires et opérationnel ainsi que sur les alliances à développé entre nos industries de défense, saluons en outre la volonté d'avancer dans ce secteur si stratégique à l'espace nos Liens sont déjà nombreux en la matière, mais nous ne devrons immanquablement, apprendre à mieux unir nos forces avec 7 autres poids lourds européens du spatial, si nous voulons faire face à une concurrence internationale de plus en plus rude, il était également important que le traité à bord de les questions migratoires qui ont été un irritant majeur ces dernières années, conduisant parfois jusqu'à la brouille diplomatique, elles ne sont pas éluder, même s'il faut bien avouer qu'elles ont traité de manière assez succinctes, retenons néanmoins qu'un mécanisme de concertation renforcée et créer au niveau ministériel et que celui-ci pourra s'appuyer sur une unité opérationnelle conjointe nos mésentente passée l'ont prouvé en Méditerranée comme dans les Alpes nous ne trouveront pas de solution efficace qui ne soit pas concerté, notre groupe restera bien sûr extrêmement attentif aux évolutions de la situation migratoire sur le terrain, mais ces nouveaux dispositifs sont, en soit, un progrès, un mot enfin sur la jeunesse, nous savons tous le rôle qu'a joué l'OFAJ dans le resserrement des Liens entre la France et l'Allemagne depuis 60 ans, ce sont près de 10 millions de jeunes qui ont pu, grâce à cette structure, participer à des programmes d'échanges, contribuant ainsi à faire de la relation franco-allemande une relation humaine et pas seulement institutionnels dans ce domaine, les échanges transalpins ne partent pas d'une page blanche, loin s'en faut, mais la création par ce traité d'un conseil franco-italien de la jeunesse et d'un service civique franco-italien viendra accélérer amplifier les contacts noués par ceux qui feront l'avenir de nos 2 pays et c'est peut-être dans la réussite de ce type de dispositif que résidera finalement le meilleur gage de succès pour le traité du Quirinal car au-delà des inévitables fluctuations de toute relation bilatérale, c'est bien le lien profond entre nos 2 peuples qui fera que ce texte résidera à l'épreuve du temps, l'expérience passée nous incite à l'optimisme : nous avons aujourd'hui l'occasion de réaffirmer solennellement et de consolider l'amitié profonde que se portent les nation française et italienne, le groupe les Républicains la saisira et soutiendra la ratification de ce traité, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à Madame Colette. Mello pour quatre minutes pour le groupe, les indépendants. Madame la présidente, madame la Ministre. Madame l'ambassadrice. Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, la France et l'Italie entretiennent une très longue relation liée à la proximité de nos 2 pays, mais aussi à notre histoire commune du temps des Gaulois et des Romains nos cultures s'influencer déjà, ensuite nous avons ensemble connu la renaissance, le palais du Luxembourg n'a, n'est-il pas un exemple cette relation et et pour ainsi dire, l'une des composantes les plus essentiels de notre civilisation nous avons fait l'Europe un peu plus tard, nous faisons partie des 6 pays fondateurs, le 25 septembre dernier Madame Giorgia Meloni a remporté les élections législatives en Italie, cette nouvelle donne politique peut paraître inquiétante, particulièrement dans le pays qui a vu naître le fascisme, l'Italie n'est cependant pas un cas isolé, d'autres élections en Europe montre la progression de l'extrémisme politique, c'est ainsi qu'en France, répartis entre gauche et droite les extrêmes sont arrivés en tête du 1er tour de la présidentielle, ils soufflent sur l'ensemble de l'Europe, un vent de radicalité chaque peuple et néanmoins souverain, le peuple italien a voté, il faut respecter le résultat de ce scrutin, cela ne nous empêche cependant pas de combattre des idées qui ont conduit à la victoire de Madame mélodies, les membres du groupe, les indépendants ont toujours lutté contre les extrémismes, nous regrettons que ce ne soit pas le cas de toutes les formations politiques de notre pays, nous sommes convaincus que l'avenir des peuples européens se trouve dans l'Union, c'est pourquoi nous sommes favorables aux initiatives qui renforce la coopération entre les États par ces coopérations, nous pouvons faire vivre nos idées et nos valeurs, la convention signée le 26 novembre 2021 avec la République italienne concerne un très grand nombre de sujets, elles resserrent la coopération de nos 2 pays dans des domaines majeurs, celui des affaires étrangères, la défense, la justice ou encore les politiques migratoires : il s'agit de sujets essentiels pour nos 2 pays, nous avons besoin de travailler ensemble pour faire avancer les choses, au-delà de ces sujets régaliens la convention concerne également l'économie et le développement durable de des priorités les plus importantes de nos pays et de nos peuples, c'est par le travail que nous pourrons améliorer la situation de nos concitoyens et de nos entreprises, cette convention ne se concentre pas seulement sur l'amélioration de l'existant, elle prépare aussi l'avenir en renforçant la coopération de nos pays, sur des sujets de pointe sur le numérique ou l'espace nous deux pays se donne les moyens de bâtir un avenir meilleur, nous serons cependant particulièrement attentifs quant aux évolutions politiques de notre voisin, la nouvelle donne politique en Italie ne correspond pas à nos valeurs, une vigilance constante s'impose, tant en matière de politique intérieure que dans les institutions européennes nous pensons cependant que ce Dan ne doit pas nous détourner de la coopération, l'Italie et la France ont besoin l'une de l'autre, en travaillant ensemble, nous pourrons faire rayonner nos idées et nos valeurs, la convention signée et tout à fait conforme à notre conviction plus d'Europe et une meilleure intégration l'ensemble des membres de notre groupe voteront donc en faveur de la ratification. La parole est maintenant à monsieur Guillaume Gontard, président du groupe Écologie Solidarité territoire pour quatre minutes. Madame Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les les rapporteurs, le groupe écologiste a demandé le retour à la procédure normale pour ce traité de coopération bilatérale entre la France et l'Italie 10 traité du Quirinal pour 2 raisons tout d'abord, il s'agit seulement du 2ème traiter de cette nature, signée par la France avec un pays européen, le précédent ça été rappelé dans le traité de l'Élysée en 1963 par le président de Gaulle et le chancelier Adenauer qui a jeté les bases du couple franco-allemand, aujourd'hui encore, malgré les tensions actuelles, moteur de la construction européenne, c'est donc un acte politique extrêmement fort que le pouvoir exécutif soumet à la ratification de notre Parlement mais le Sénat se prononce sur la ratification de ce traité, signé par le président Macron et Draghi alors que l'Italie est à un tournant politique de son histoire et vous en avez curieusement peu parler, Madame la Ministre, tournant politique avec la victoire de la coalition d'extrême droite et de droite qui a permis l'accession à la présidence du Conseil de la dirigeante fasciste Giorgia Meloni cette victoire de l'extrême droite dans un pays fondateur de l'Union européenne est un moment d'une gravité extrême qui doit interpeller tous les républicains que nous sommes, c'est, disons-le clairement, en grande partie le résultat d'un échec de la politique communautaire, l'échec d'abord des politiques d'austérité qui ont prévalu après la crise économique de 2008 et qui ont considérablement appauvrie et affaiblie, les pays du sud de l'Europe, l'échec ensuite de notre politique migratoire des règlements de Dublin Dublin II et Dublin III qui, en refusant le droit de libre installation des personnes migrantes et en forçant l'enregistrement des demandes d'asile dans le 1er pays européen visiter ont abandonné les pays méditerranéens l'Italie au 1er chef face au défi migratoire. Nexign auront cependant pas les dirigeants italiens, au prix en en 1er rang desquels le triste sire Berlusconi de leurs responsabilités, mais reconnaissons, celle de la France et de l'Union européenne, l'ironie, c'est que si nous avions conclu et appliquer ce traité du Quirinal, il y a 20 ans, nous aurions sans doute éviter l'Italie de sombrer dans l'abîme fasciste, il s'agit des ambitions portées en matière de souveraineté économique, notamment industriels ou pour et je cite une politique européenne de migration et d'asile et des politiques d'intégration fondée sur les principes de responsabilité et de solidarité partagée entre les États et prenant pleinement en compte la particularité des flux migratoires alors frontières respectives, les dispositions de ce traité et notamment la construction d'un réflexe franco-italiens sont de nature à permettre à Rome de sortir de son relatif isolement sur la scène européenne, nous avons bien conscience que prolonger isolement du gouvernement italien Nandi aura en rien la montée du nationalisme et de l'euroscepticisme qui ont permis la victoire de l'extrême droite, nous ne voulons pas rejeter ce traité qui porte en lui une ambition historique pour l'amitié franco-italienne, mais aujourd'hui, alors que les héritiers de Mussolini ont pris le pouvoir le préalable à toute coopération franco- italienne renforcée doit être d'une intransigeance absolue sur le respect de la démocratie, le respect des droits fondamentaux, notamment le droit des femmes et des minorités aussi, Madame la Ministre, nous vous demandons des garanties et précision qui me semble nécessaire après votre intervention, la France suspendra-t-elle l'application du traité quand ces droits seront bafoués refusera-t-elle de remettre à la justice italienne des militants antifascistes qui victimes de répression politique se réfugieraient sur son sol soit organisé chaque année un sommet intergouvernemental avec un pouvoir fasciste veut-elle poursuivent la normalisation de l'extrême droite, que le président de la République semble avoir entamé dimanche soir, ce traité est historique, sa portée, je l'ai dit symbolique et exceptionnel aussi, au regard du contexte politique actuel, nous avons besoin de garanties fermes du gouvernement pour nous prononcer en faveur de sa ratification à défaut nous serons contraints de nous abstenir merci. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est non sans émotion que je prend aujourd'hui la parole pour exprimer la totale adhésion du groupe RDPI à ce traité franco-italien de coopération déjà ratifié par les 2 chambres italienne ainsi que par l'Assemblée nationale en juillet dernier une émotion personnelle néanmoins partagé par nombre d'entre nous ici, qui avant des ascendances transalpines et qui vivons avec amertume les montagnes russes qui trop souvent régissent les relations entre nos 2 pays et parfois entre nos 2 peuples, mais 2 grands-pères ont quitté l'Italie il y a près d'un siècle pour fuir le fascisme, ils se sont vite intégrés et ont trouvé épouse ici en France et ont choisi de ne pas à prendre la langue de Dante à leurs enfants l'Italie est longtemps resté une blessure familiale et lorsque j'ai voulu étudier Netanyahu qu'au collège, ma mère a décrété que non, ce serait l'allemand, la langue, selon elle, des bons élèves c'est un adulte que j'ai finalement découvert le pays de mes aïeux, sa culture, sa langue, allant jusqu'à adhérer à cet OVNI politique et le Partito radical de feu Marco panel concrètement c'est par le bi-culturalisme qui s'est invitée en moi, que j'ai véritablement saisi l'enjeu fondamental de la construction européenne, j'ai compris que l'Union européenne pour formidable avancée qu'elle fut, et elle de morts ne pouvait tout leviers les plus essentiels pour bâtir un authentique vivre ensemble européen, j'entends par là, la culture, l'action les l'éducation et l'agir politique de Muray des compétences de nature nationale et donc troupes partagé entre États membres, en faveur de l'enseignement et de la culture qui pèse en moyenne plus de 5 pour 100 de nos PIB nationaux respectifs ne représentent qu'à peine 1 virgule 4 pour 100 du budget global de l'Union européenne qui lui même, rappelons-le, n'équivaut qu'à un peu plus de 1 % du PIB de l'Europe se vivre européens ne se décrète pas, et on peut vivre parfois sous le même toit européen et ne pas s'aimer, c'est le cas, quand nous ne voyons pas ce que l'autre tient de nous en lui et ce que nous tenons de lui en nous au delà des guerres et des rivalités qui nous ont déchiré, il est urgent aujourd'hui de retrouver les filles l'ont souvent oublié de notre histoire et de notre culture commune pour construire ensemble un destin partagé après les horreurs du nazisme et de la seconde guerre mondiale : la réconciliation franco-allemande a été le plus important défi de l'Europe des décennies, des décennies qui suivirent ce qui paraissait impensable impensable en 1945 c'est bel et bien réalisé sans cette réconciliation jamais la réunification allemande et l'ouverture de l'Union à son flanc Est Nur possible le traité de l'Élysée de 1963 instaurant une coopération renforcée en matière de diplomatie, de jeunesse et de culture, a joué un rôle majeur dans ce processus de rapprochement avec l'Allemagne, il est clair que nous deviendrons que trop attendu pour avoir une approche similaire avec l'Italie, notre second partenaire économique et surtout le pays avec lequel notre filiation historique et culturel et la plus ancienne et la plus intense à est à l'heure où la guerre sévit à nouveau en Europe que les relations internationales se brutalise et devient impératif d'apaiser nos querelles de cousinage et de voisinage, de raviver les Liens qui nous rassemble le traité qui nous est aujourd'hui proposé bien plus ambitieux que celui de l'Élysée dans les domaines de coopération envisagée sont plus vaste et plus nombreux, bien sûr, sa mise en oeuvre effective apportera davantage que le symbole de sa ratification est certes l'Italie vient de se doter d'un gouvernement dont la principale composante sur la télé d'Italia est la seule formation qui s'est opposé à sa ratification mais le réalisme, plus encore que l'optimisme me conduit à penser que c'est une chose que d'avoir une posture dans l'opposition et que c'en est une autre, lorsqu'on se trouve en responsabilité, je vous remercie. La parole est maintenant Monsieur André Vallini pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, et ce pour 7 minutes. Chère madame la présidente, madame la ministre, madame l'ambassadrice, mes chers collègues, j'ai été touché par les paroles de notre collègue Gattolin je partage avec lui des origines italiennes, ne l'aurais pas son lyrisme, j'en serais bien incapable, pour dire à quel point ce moment est important pour la très nombreuse communauté française d'origine italienne. Alors l'inconvénient de parler en dernier ou en avant-dernier, chers collègues, c'est que tout a été dit, ou à peu près sur le contenu du traité aussi bien sûr ce son contenu interne, si j'ose dire bilatéral que sur son contenu européen, donc je vais écourter mon propos pour me concentrer sur la question qui nous occupe tous ce soir donc, vous avez tous parlé, que va-t-il advenir de ce traité dans les mois et les années qui viennent. Il peut rester un simple parchemin lettre morte sans aucune conséquence, soit l'inverse, il peut servir et c'est ce que nous souhaitons bien sûr de tremplin à une véritable coopération approfondie entre nos 2 pays cet événement, cette dernière hypothèse, qu'il faut souhaiter, et qu'il nous faudra favoriser. ça a été dit aussi avant moi, la France et l'Italie sont les deuxièmes partenaires commerciaux, la France et le de la 2ème destination des étudiants italiens en mobilité à l'étranger, et la France est le 2ème, pays d'origine des étudiants en mobilité en Italie. Le MEDEF et le patronat italien, ont des Liens très étroits, hé bien sûr nos relations culturelles, universitaires sont très intense. Alors bien sûr, la droite, la droite, ils n'ont pas l'extrême droite, parce qu'en Italie, la droite, c'est l'extrême droite en France. Et la droite française, c'est le centre-droit en l'Italie donc la droite italienne a gagné les élections et elle ne s'est guère montré francophile, jusque là, ça a été rappelé avant moi, le parti de madame Meloni Fratelli d'Italia a voté contre ce traité. La Ligue aussi a voté contre, considérant qu'il servait avant tout les intérêts français des sondages d'ailleurs de façon plus générale et il faut en avoir conscience des sondages montrent que près de 40 pour 100 des Italiens ont de l'antipathie pour la France de l'antipathie parce qu'il nous reproche notre suffisance, entre guillemets, c'est eux qui le disent, ce n'est pas moi notre arrogance parfois. C'est d'ailleurs un sentiment partagé par d'autres peuples européens, il faut aussi le savoir. D'ailleurs, il suffit de regarder le traitement médiatique qui a été réservé des 2 côtés des Alpes au traité du Quirinal, on en a beaucoup parlé en Italie comme d'un événement très important, on en a à peine parler en France 20 secondes au journal de 20 heures et encore. Alors que va faire ce le goût, le nouveau gouvernement italien de ce traité, on entend souvent le terme de post-fasciste, j'ai même entendu fasciste dans la bouche de mon prédécesseur Gontard pour décrire madame Meloni, c'est un peu rapide certes sa trajectoire s'inscrit dans l'histoire du mouvement néofasciste, le MSI italien et une partie de son entourage, c'est vrai, et de ses électeurs, c'est vrai aussi, revendique la filiation mussolinienne, c'est vrai, à commencer par le président du Sénat, il n'y a Tio Benito La Rousseau. Mais il est faux de dire qu'elle a imposé que madame Meloni a imposé sa domination sur la droite italienne en proposant 100 après une sorte de nouvelle marche sur Rome, ce qu'elle a réussi, en fait, et je parle en ayant lu comme vous, beaucoup de de chroniques de tribune, j'ai déjeuné encore hier avec Marc Lazar, qui est l'un des meilleurs spécialistes actuels de l'Italie contemporaine, ce qu'elle a réussi, madame Meloni c'est une sorte de synthèse entre le cadre géopolitique de l'Alliance Atlantique, le cadre économique de l'Union européenne et des valeurs très conservatrice sur le plan sociétal, notamment par rapport à l'avortement par rapport aux minorités à la communauté LGBT etc donc c'est une opération compliquée qu'elle a réussi. Pour se recentrer et rassurer les milieux économiques et financiers à laquelle elle s'est livrée et à la rassurer aussi les alliés de l'Italie, et a même fait une vidéo en français pour rassurer la France pendant la campagne électorale, elle a même déclaré, mon gouvernement a une ligne étrangères clair, je la cite : l'Italie est pleinement et la tête haute dans l'Union européenne et dans l'OTAN, j'ajoute que, hier, lors de sa déclaration de politique générale devant le Parlement italien, elle a abjuré le fascisme. Et elle a abjuré notamment et heureusement les lois raciales de 1938 pour autant va-t-elle réaffirmé la prééminence des nations et de leur souveraineté à rebours de l'européisme et c'est positif dans ma bouche, de l'européisme italien traditionnel. Va-t-elle emprunter la voix polonaise ou la voix hongroise regard notamment des valeurs européennes, ce sera le cas échéant, ce serait le cas échéant à la Commission européenne et au Parlement européen de le constater et d'y répondre. En tout cas à ce jour, il faut noter qu'elle a nommé à des postes clés des personnalités qui situe son gouvernement dans une continuité européenne internationale notamment Antonio Taya Annie aux Affaires étrangères, ancien président du Parlement européen Georgetti au ministère de l'économie, il était déjà ministre de Mario Draghi. J'ajoute que son gouvernement n'est pas sûr de durer aussi longtemps qu'il le souhaiterait sa majorité composite tiraillée entre les berlusconiens, d'un côté et la Ligue du nord, de l'autre, en tout cas le peuple italien a voté, ça a été dit avant moi, il faut prendre acte de son choix et éviter, Madame la Ministre, permettez-moi de relever cette maladresse, éviter les jugements hâtifs sur ce choix, sauf à nous retrouver taxer à nouveau d'arrogance : vous avez une déclaration pour le moins mal à droite, il y a quelques jours, elle a été ressentie comme telle. Depuis longtemps, l'Italie, comprend mal notre relation privilégiée avec l'Allemagne, estimant en être injustement exclu, je termine, madame la présidente. Alors saisissons l'occasion de donner un un autre relation avec l'Italie, l'importance qu'elle mérite, c'est à l'échelle du temps long qu'un truc, un traité peut se se juger se juger donnant du temps au temps, donnons du temps à se traiter le groupe socialiste votera ce traité historique et pour ma part, je le ferais avec enthousiasme, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à la présidente : Éliane Assassi, présidente du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

Madame la présidente, madame la ministre, madame l'ambassadrice, mes chers collègues, ce traité de coopération renforcée entre notre pays et l'Italie, signé, donc le 26 novembre 2021 et que nous examinions aujourd'hui contient plusieurs mesures qui majoritairement recueille notre approbation, mais comme je me plais souvent à le dire, il y a le texte. Et le contexte et nous ne pouvons donc ignorer ici les résultats des récentes élections italiennes bien après donc le vote unanime à l'Assemblée nationale, la devise de l'Europe unie dans la diversité est une belle devise mais elle risque d'être malmené avec l'arrivée au pouvoir en Italie d'une coalition de droite au sein de laquelle on trouve les Frères d'Italie partie pas de droite, à parti d'extrême droite, issu de la mouvance post-fasciste, la présidente de ce parti Madame Giorgia Meloni est aujourd'hui la première ministre italienne et cela n'augure rien de bon à notre sens, on ne peut donc ignorer cette situation est fort et faire comme si ce serait un moment un mauvais moment à passer non. La situation est grave parmi les nombreuses mesures de ce traité de coopération bilatérale renforcée figure un durcissement des règles migratoires entre nos 2 pays, or madame Meloni milite en faveur d'une politique migratoire très strict et plaide pour la fin : la fermeture des ports afin d'empêcher les navires d'ONG, de débarquer les migrants, elle entend par ailleurs multiplié les centres de surveillance et les expulsions à titre d'exemple, en août 2019, elle a fait la démonstration d'une rigidité glaciale alors que le navire de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, transportait 147 migrants à son bord, les partis politiques italiens se sont déchirés sur leur accueil en Italie face à cela, madame Meloni avait proposé une réponse inquiétante : celle de créer un blocus Naval qui empêcherait l'embarquement des migrants depuis la Libye ou la Tunisie, de plus, le traité présente une source d'inquiétude supplémentaire : la coopération pour une politique migratoire est appréhender sous un prisme répressive répressif en effet, ce traité n'envisage aucune, aucune proposition pour organiser des opérations de sauvetage conjoint des migrants comme l'opération Marée Nostrum lancé après le drame de lampes et 12 cette vision conduit à des situations dramatiques ainsi depuis plusieurs années, on ne compte plus le nombre de migrants morts en Méditerranée, devenu un véritable cimetière le rapport de l'Agence de l'ONU pour les migrations répertorie 2836 décès et disparitions en Méditerranée centrale depuis 2021 et nous craignons que les positions de la nouvelle Première ministre ne fasse qu'agrandir cet enfer, les choix politiques anti-immigration porté par madame Meloni ne rendent pas hommage à l'histoire à celle de l'Italie à la richesse et à la diversité de la culture et des cultures et à l'apport de cette diversité pour le rayonnement de ce pays, comme je l'ai précisé ce traité de coopération entre nos 2 pays et je dirais surtout, surtout entre nos 2 peuples est acceptable sur beaucoup de mesures mais comment ignorer cette épée de Damoclès qui plane sur le devenir de celles et ceux qui quittent leur pays pour fuir la guerre, la famine, le réchauffement climatique, l'atteinte à la dignité humaine, le choix de madame Meloni ne tend pas la main. Une main ouverte des yeux attentifs, une vie la vie à se partager, comme l'écrivait Paul Éluard par amitié pour le peuple d'Italie et les Liens forts qui nous unissent, nous ne voterons pas contre ce texte mais nous nous abstiendrons. Madame le Ministre, je sais que vous avez demandé reprend la parole, mais le président bon aussi souhaite s'exprimer si vous êtes d'accord, je donne la parole dès maintenant. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je veux simplement ramener ce débat à sa juste mesure je rappelle 2 ou 3 choses : tout d'abord, c'est les traités sont signés entre les peuples, entre les pays et donc ce n'est pas avec le gouvernement qui est issu du reste d'élections libres, qui vient d'avoir lieu en Italie que ce traité est proposé à notre ratification je rappelle qu'il a été préparé par l'ancien gouvernement de monsieur Draghi et donc ces dispositions s'impose au gouvernement français comme ils imposent au gouvernement italien, il reviendrait au nouveau gouvernement italien, le cas échéant de le dénoncer, mais elle n'est pas le cas et on ne peut suspecter, pour l'instant, les intentions de ce gouvernement, laissons la chance à un gouvernement démocratiquement élu, par ailleurs, je rappelle combien nous avons besoin de renforcer et d'approfondir cette relation avec l'Italie qui, à bien des égards, et singulièrement mes, mes collègues de la commission des affaires étrangères et la défense qui débattent régulièrement avec moi et avec nous, les personnalités qui nous rendent visite des problématiques de la Méditerranée ça bien combien les sujets de défense se repose notamment sur la France, l'Italie, l'Espagne, des pays qui sont un petit peu responsable de la situation dans cette région du monde, donc je crois qu'il faut franchement donné cette chance à ce à ce traité, l'Italie est un grand pays tant de Liens historiques d'histoire, de culture, de civilisation d'économie nous relie et puis de défense aussi, donc moi je souhaite vivement que nous ayons de la part du sénat une réponse très franches pour approuver et donner cette chance à cet approfondissement de la relation amicale entre la France et l'Italie, et je souhaite que l'ambassadrice, dont c'est la nouvelle la première apparition au Sénat ne soit pas déçu par la sagesse des sénateurs merci.

du sénateur Gattolin et de nombreuses autres sénateurs en faveur du peuple italien, je vais répondre à quelques questions, messieurs les sénateurs Gontard je je vous laisse la responsabilité du qualificatif que vous avez utilisé ce que je note c'est que madame Meloni dans son discours de politique générale devant la Chambre italienne s'est exprimé elles-mêmes sur son rapport à l'histoire de l'Italie et qu'elle a dit que le fascisme avait constitué le point le plus bas de cette histoire, alors cela ne signifie pas que nous partageons la ligne politique du gouvernement italien, ce sont même 2 offres politiques très différentes que nous porterons dans la perspective notamment des élections européennes de 2024 et c'est un combat politique légitime et qu'il faudra avoir de manière respectueuse de nos démocraties et de nos électeurs et électrices, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit avec ce traité, madame la sénatrice, laissez-moi parler, je vous prie, écoutez, madame la sénatrice, d'une part je vous ai laissé parler moi aussi, je crois, monsieur le du coup j'en ai perdu mon monsieur le président, monsieur le rapporteur, comme la sénatrice Mélo ont très bien défini ce qu'il y a dans ce traité ce traité, c'est une structure et c'est une matrice et il sera ce que nos 2 peuples en feront, et là il y a plein de collaboration possible, je dis bien possible, à nous de saisir ou non les opportunités dans le domaine économique, dans le domaine automobile par exemple, nous avons Stellantis en commun dans le domaine des microprocesseurs nous avons STM micro économique qui va bientôt une ouvrir une usine en France à Crolles près de Grenoble, nous avons des intérêts de défense conjoint, certains d'entre vous l'ont souligné à la fois en termes de de frontière méridionale et en terme de synergies de pardon de synergies opérationnelles pour des opérations extérieures, et je pense à il il y a des coopérations industrielles pour l'espace, à la fois institutionnelle et effective institutionnel, vous pouvez penser à nos travaux conjoints au sein de l'Agence spatiale européenne, il y a surtout, et je crois que c'est le plus important, une des choses les plus importantes, le rapprochement des jeunes Français avec les jeunes italiens, parce que c'est cela qui fera l'amitié dans nos pays et c'est cela qui fera une union forte et démocratique et donc là il y a les services civiques, il y a toutes les mobilités qui ont été notés, il y a la coopération transfrontalière, qui je crois est l'expression même de l'amitié et aussi parfois des difficultés qu'il y a à mettre en oeuvre l'Union européenne, messieurs les et mesdames les sénateurs, la question des migrations a été soulevée, je rappelle que la migration, nous avons avancé avec le pacte Asile migration dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, il y a, il y a 2 mots responsabilité et solidarité, responsabilité dans l'accueil des migrants qui trop, comme très souvent arrivent en Italie et solidarité de la part de pays où les flux sont secondaires comme la France, en conclusion, je voudrais vous remercier pour ces débats qui était riche intéressant et l'expression de l'amitié entre nos 2 peuples, et je vous souhaite un bon vote merci. nous passons à la discussion de l'article unique, hein, que je vais mettre aux voix quand j'aurais mis aux voix l'article unique qui constitue l'ensemble du projet de loi, le vote sur cet article vaudra vote sur l'ensemble du projet de loi il y a une demande d'explication de vote de Monsieur Tabarot, il y a-t-il, y aura-t-il d'autres demandes d'explications de vote Monsieur Tabarot, vous avez la parole. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, je voterai ce traité car je souhaite que la France n'auront pas ses Liens avec notre voisin, il ne se cachent pour rencontrer les autorités italiennes, les 2 soeurs latines semble acté les voies d'une d'un apaisement constructif qui ouvrent de nombreux chemins de coopération et je souhaite que cela continue, avec notre partenaire européen parmi ces pistes, la coopération transfrontalière occupe une place remarquée, on notera avec intérêt la mention de service public communs en matière de transport routier et ferroviaire, il y a le plus illustre le Lyon-Turin mais il y a aussi la ligne de chemin de fer Cuneo Vintimille qui traverse la France et le tunnel routier de Tende 2 infrastructures transfrontalières, particulièrement touchée par la tempête Alex, j'attire votre vigilance sur l'impérieux besoin de rehaussement et d'accélération de modernisation de ces 2 infrastructures les 2 États doivent s'y employer, aux côtés des collectivités mais également sur l'appel que je lance à ne pas être candide ce traité consacrent des instances de dialogue politique bilatérale qui existe déjà et depuis longtemps, comme les CIG qui n'ont vraiment pas donné encore toutes les réponses satisfaisantes et je pense à la révision de la convention d'exploitation de la ligne de 1970 la nouvelle instance créée par le traité dit comité de coopération frontalière pourrait aspirer à n'être qu'un paravent bureaucratique, s'il ne se part pas d'une impulsion politique qui permettrait de lever certains obstacles vitaminé par le traité du Quirinal j'accorde à cet accord franco-italien satisfecit mais à la condition qu'il soit vraiment fécond, notamment sur la question qui me concerne plus particulièrement dans cet hémicycle, celle des transports, un vrai Return du couple franco-italien ou une coquille vide, je suis un éternel optimiste et je veux y croire. Merci madame la présidente, c'est pour les écologistes, un vote compliqué vous savez que les écologistes sont depuis toujours profondément pro-européen profondément fédéraliste et que l'intensification de la collaboration entre les pays membres et entre les peuples et pour nous un élément fondamental de la construction européenne et de l'Inde, l'intensification du projet européen dans son ensemble, nous savons aussi que ce traité est là pour pour durer pour j'espère plus longtemps que le gouvernement italien actuel, et que il devrait évidemment lui lui survivre et et se dérouler dans des circonstances qui ne sont pas les circonstances actuelles, néanmoins, il se déroule dans un contexte c'est ce contexte c'est à la fois la montée de l'extrême droite dans un certain nombre de pays, je note que que mon collègue considère qu'il n'y a visiblement pas d'extrême droite en Italie je considère pour ma part que Georgia Meloni est effectivement une dirigeante néo-fasciste et je, je, je me sens parfaitement responsable de mes propos, c'est un contexte et nous ce dont nous avons besoin, l'Assemblée nationale la ratifié dans un moment qui était avant les élections, voilà, il s'est passé quelque quelque chose cet été le gouvernement de Draghi est tombé un autre gouvernement lui a succédé, c'est un gouvernement qui porte des valeurs qui sont à l'opposé total à la fois des nôtres, mais aussi de l'Union européenne dans son ensemble et la question que nous avons c'est qu'est-ce que le gouvernement va faire au moment où les droits et libertés fondamentales seraient, je ne sais pas, j'espère que ce sera pas le cas seraient menacés en Italie, comment comptez-vous appliquer ce traité, quelles sont les garanties dans l'application de ce traité, au moment où on commence à avoir des violations des droits et libertés fondamentales, je crois que Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu à ce sujet, j'ai pas bien compris si on allait dans le cas où l'Italie prenait le chemin que j'espère, ne prendra pas comment on collabore avant les conseils des ministres à ce qu'on va vraiment coordonner nos positions, c'est pour l'instant des questions auxquelles nous n'avons pas eu les réponses je le regrette, si vous les avez, vous pouvez toujours nous apporter, mais sans les avoir, nous serons contraints de nous abstenir. Sur le président, Marseille. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, je voudrais dire que tant que président de la du du groupe d'amitié France-Italie ici au Sénat, que je fais miennes les propos tenus par le président Cambon, je crois qu'il est important, au-delà des gouvernements, c'est fait pour ça, les traiter au-delà des dirigeants qui sont élus démocratiquement et nous n'avons pas à nous immiscer dans les choix des autres pays, sinon on va faire une Europe on ne parlera plus. On ne parlera plus. Avec les Polonais, on ne parlera plus avec les Hongrois, on ne parlera plus avec les Suédois, on ne parlera plus que les Autrichiens, j'imagine qu'il va falloir changer de dimension, les salles de réunion européenne pour nous réunir, de plus en plus dans des cabines téléphoniques ou des petites salles appropriées, je crois qu'il ne nous appartient pas, on peut avoir des des opinions peut avoir des sensibilités, c'est légitime, on peut les exprimer, c'est fait pour ça, mais les traiter, c'est fait pour durer, et ce qui est important, c'est la relation entre la France et l'Italie, ça n'est pas le problème des relations entre un gouvernement et un autre ces gouvernement il bouge, ça a été dit, ça a été dit par les uns ou par les autres, ça peut même aller parfois très vite, bon nous avons nous même une situation qui n'est pas la plus formidable qui soit bon et donc je ne crois pas qu'il nous appartient de donner des leçons, et je pense que il est important, comme cela a été dit en particulier par le rapporteur et par le président bon que nous puissions marquer ce qui fait le lien très fort entre la France et l'Italie durablement à travers les années, c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous travaillons ici au Sénat avec le groupe d'amitié avec nos amis italiens qui au demeurant n'ont qu'un groupe d'amitié, il y a pas un groupe d'amitié Sénat un groupe d'amitié, assemblée nationale il y a un seul groupe d'amitié pour les 2 assemblées et c'est la raison pour laquelle, comme l'a souligné la ministre et plusieurs orateurs également le travail parlementaire est important car ce travail parlementaire, il a permis au moment des crises au moment des crises de continuer à agir justement pour maintenir ce lien et exprimer nos points de vue et essayer de faire évoluer les situations et c'est la raison pour laquelle évidemment une nouvelle fois, j'appelle à voter ce traité. Merci madame Merci madame la présidente, madame la sénatrice, vous connaissez les valeurs que nous portons et je crois que vous les partagez vous connaissez aussi les valeurs que porte l'Union européenne, le cadre légal et réglementaire de l'Union européenne avec un état de droit qui s'applique à nous tous, y compris d'ailleurs la France, je ne vais pas spéculer sur les actions du gouvernement, je n'ai pas mon rôle et ce n'est pas notre rôle, je crois ce que je vous rappelle, c'est que ce traité, il sera ce que l'on fait ces termes traité d'amitié entre 2 peuples, il est à construire, merci. Bien comme il n'y a plus d'explications de vote, à ma connaissance, je vais donc mettre aux voix l'article unique constitue ensemble de le projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Le projet de loi et donc adopté définitivement mèches. Mes chers collègues. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 30 pour la déclaration du gouvernement, en application de l'article 50 tirer hein la Constitution relatives à la guerre en Ukraine et aux conséquences pour la France, la séance est suspendue.